La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, améliorant l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale

plus lisible et plus efficace. Nombre de territoires sont aujourd'hui marqués par la petite délinquance, qui altère la tranquillité publique, dégrade les conditions de vie et donne le sentiment d'une impunité faute d'une réponse judiciaire rapide et immédiatement visible. Les dégradations, les insultes, les rodéos urbains et les petits trafics en tous genres affectent le quotidien des Français et génèrent leur exaspération. Afin de lutter contre ces incivilités et ce sentiment d'impuissance chez les victimes, le Gouvernement s'est engagé dans une politique visant à renforcer la justice de proximité. Le Premier ministre l'a rappelé lors de son discours de politique générale : les Français veulent une justice au coeur des territoires, des villes et de leurs quartiers. Elle doit être rendue au plus près de nos concitoyens. La réponse à ce besoin de protection et de sécurité passe d'abord par des moyens supplémentaires. Le budget important que j'ai décidé de consacrer au renforcement de la justice de proximité est à la hauteur des enjeux. Les frais de justice ont été augmentés de 127 millions d'euros. Ils permettront notamment de mobiliser davantage les délégués du procureur, qui sont au plus près des justiciables et des victimes. 13 millions d'euros permettra de recourir plus largement à des magistrats honoraires et à des magistrats à titre temporaire et 20 millions d'euros seront investis au profit du milieu associatif de la protection judiciaire de la jeunesse, pour renforcer la prise en charge rapide des délits du quotidien. Enfin,

Mais la justice de proximité passe également par une politique pénale qui prend en compte les litiges de basse intensité et qui accompagne nos concitoyens les plus démunis. Dans une circulaire de politique générale du 15 décembre 2020, j'ai décliné les actions que je souhaitais voir rapidement mises en oeuvre pour faciliter l'accès au service public de la justice et apporter une réponse pénale crédible, effective et rapide qui prenne en compte les victimes, bien sûr, tout en assurant la réinsertion des auteurs. J'ai demandé un renforcement des audiences foraines et des permanences dans les lieux d'accès au droit, aujourd'hui appelés « points justice ». Je souhaite tout particulièrement accroître le périmètre d'intervention des délégués du procureur, qui font un travail indispensable et qui apportent, en lien étroit avec les parquets, une réponse pénale de proximité et de grande qualité. J'ai demandé aux procureurs de la République de veiller à leur forte mobilisation sur l'ensemble du territoire, afin d'être plus proche de nos concitoyens. J'ai d'ailleurs pris, le 21 décembre 2020, un décret qui précise les missions des délégués et leur donne la possibilité, pour l'exercice de leurs missions, de tenir des permanences délocalisées. L'autorité judiciaire doit par ailleurs être plus réactive face aux incivilités. De sa rapidité dépend l'efficacité de son action. J'ai souhaité que les parquets maîtrisent davantage les délais de réponse pénale et qu'ils créent, dans les services d'une certaine importance, des filières dédiées au traitement des infractions du quotidien. La justice doit également être plus proche des acteurs locaux, en réaffirmant des relations partenariales avec les collectivités, les élus, le tissu associatif et les acteurs de terrain, pour apporter des réponses plus réactives face aux incivilités. L'amélioration de la justice de proximité passe enfin par des dispositions pénales plus efficaces pour lutter contre la petite délinquance qui parasite la vie de nos concitoyens. Pour les délits de faible gravité, il faut des réponses rapides et constructives. C'est l'objet de la proposition de loi que vous examinez.

pour objet de favoriser, dans le cadre d'une transaction, le recours au travail non rémunéré par les maires face aux incivilités commises sur leurs communes. Il s'agit là d'une belle avancée ; j'y suis, à ce titre, très favorable. Cette proposition de loi simplifie par ailleurs les modalités d'exécution du travail d'intérêt général (TIG). Ce volet est essentiel, car cette réponse pénale, très pédagogique, n'a de sens que si elle est rapide. Or, aujourd'hui, le délai moyen d'exécution d'un TIG est de quatorze mois, ce qui est incompréhensible et totalement inefficace. Nous disposons de vingt mille postes de travail d'intérêt général et nous continuons à les développer. Nous avons des lieux d'accueil et des référents dans les collectivités. Il nous faut maintenant réduire impérativement le délai d'exécution de cette peine. La déjudiciarisation et la simplification des modalités de mise en oeuvre du TIG, que nous soutenons, vont largement y contribuer. Ce texte complète par ailleurs les mesures alternatives aux poursuites déjà prévues par le code de procédure pénale. Le procureur de la République pourra ainsi demander au délinquant de remettre en état les lieux ou les objets dégradés, ou le contraindre à verser une contribution citoyenne à une association d'aide aux victimes. Ces sanctions à la fois punitives et éducatives vont dans le bon sens. S'agissant notamment des jeunes ou des primo-délinquants, elles sont les mieux à même de prévenir la récidive. La justice de proximité doit répondre au défi de réconcilier la justice du quotidien avec ses usagers. Un budget important, une politique pénale adaptée aux territoires, des dispositions plus efficaces : voilà la justice qui protège ! La proposition de loi que vous examinez y participe significativement, en renforçant la proximité, l'efficacité et la rapidité de la réponse pénale. Le Gouvernement

afin de les aider à rendre la justice au plus près de nos concitoyens et à répondre sans délai aux petits délits du quotidien. Elle répond ainsi aux objectifs que le Premier ministre Jean Castex avait assignés au ministère de la justice dans son discours de politique générale. Cette proposition de loi fait suite à une circulaire de la chancellerie, en date du 15 décembre 2020, qui incite les chefs de juridiction à prendre différentes initiatives pour se rapprocher du terrain, tout en prenant mieux en charge les victimes. En allouant des moyens nouveaux au recrutement de magistrats à titre temporaire, de magistrats honoraires ou de délégués du procureur, le budget de la justice devrait faciliter la mise en oeuvre de ces mesures. Le texte dont nous sommes saisis résulte d'une initiative parlementaire, puisqu'il a été déposé par nos collègues députés du groupe Agir ensemble. Il présente néanmoins un caractère assez technique et plusieurs dispositions qu'il contient sont très ponctuelles. des dispositions de quatre catégories : des mesures qui concernent les alternatives aux poursuites et la composition pénale ; la mise en oeuvre des peines de travail d'intérêt général le recouvrement des contraventions ; enfin, des mesures de simplification des procédures concernant l'appel des jugements d'assises et les pourvois en cassation. Sur le premier volet, relatif aux alternatives aux poursuites et à la composition pénale, rappelons que ces deux procédures sont mises en oeuvre par le parquet dans le but d'apporter une réponse pénale à des infractions de faible ou de moyenne gravité sans passer par une juridiction de jugement, ce qui évite d'engorger les tribunaux. représentent aujourd'hui une part considérable de l'activité des parquets, de l'ordre de 40 %. La composition pénale est entourée d'un plus grand formalisme, puisqu'elle est soumise, sauf exception, à la validation d'un juge du siège. proposition de loi complète et précise la liste des mesures pouvant être mises en oeuvre par le parquet. Concernant les alternatives aux poursuites, elle précise que l'auteur des faits pourra être amené à se dessaisir au profit de l'État de biens qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit. Elle introduit également des interdictions d'entrer en contact avec la victime ou avec des complices. Elle crée enfin- c'est sans doute la mesure la plus innovante -une contribution citoyenne, d'un montant maximal de 3 000 euros, que l'auteur des faits serait obligé de verser à une association d'aide aux victimes.

tout en exprimant une forme de reconnaissance pour le travail remarquable accompli par ces associations auprès des victimes d'infractions. Concernant la composition pénale, le texte prévoit de porter de soixante à cent le nombre maximal d'heures de travail non rémunéré (TNR) pouvant être effectuées et il ouvre la possibilité de suivre un stage de responsabilité parentale. Il prévoit également de supprimer l'obligation de validation par un juge du siège des compositions conclues en matière contraventionnelle. En ce qui concerne le travail non rémunéré, la commission a adopté un amendement afin de l'inclure dans le champ de l'expérimentation prévue par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Cette expérimentation vise à évaluer dans quelle mesure le secteur de l'économie sociale et solidaire peut participer à l'accueil des personnes condamnées à une peine de travail d'intérêt général. Il nous paraît intéressant que le secteur de l'économie sociale et solidaire puisse, lui aussi, accueillir des travaux non rémunérés. Au moment de dresser le bilan de l'expérimentation, il serait ainsi possible de croiser le regard du parquet et celui du juge de l'application des peines afin de disposer d'une évaluation plus complète. Je remercie le Gouvernement d'avoir accueilli favorablement notre suggestion de modifier le code de la sécurité sociale afin que les personnes qui effectuent un travail non rémunéré dans le cadre d'une transaction conclue avec le maire puissent être indemnisées en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Cette modification permettra de combler une lacune qui compliquait la vie de nos communes. Sur une proposition d'Alain Richard et d'autres collègues du groupe RDPI, la commission a également souhaité autoriser l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) à mettre des biens immobiliers saisis dans le cadre d'une procédure pénale à la disposition d'associations ou de fondations reconnues d'utilité publique ou d'organismes participant à la politique du logement.

Le deuxième volet du texte vise à fluidifier l'exécution des peines de travail d'intérêt général (TIG). Ces dernières présentent un réel intérêt pour prévenir la récidive et favoriser la réinsertion sociale et professionnelle des condamnés. L'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice (Atigip) a été créée à la fin de l'année 2018 pour prospecter de manière plus systématique les employeurs susceptibles de proposer des TIG. Deux mesures complémentaires sont envisagées par le texte. Premièrement, il est proposé de confier aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) certaines tâches actuellement dévolues au juge de l'application des peines les directeurs de SPIP deviendraient compétents pour fixer les modalités d'exécution de la peine et seraient chargés d'instruire les demandes des employeurs désireux de proposer des TIG. Responsable de la bonne exécution des peines, le JAP conserverait toutefois la possibilité de statuer lui-même, lorsque cela lui paraît justifié. Dans une large mesure, ces dispositions ne font qu'entériner la pratique constatée sur le terrain : dans les faits, c'est bien le directeur du SPIP qui assume ces missions, tandis que le JAP se contente, sauf exception, de valider les décisions qui lui sont soumises.

Sur ce volet du texte, la commission s'est surtout attachée à clarifier les interventions respectives du directeur du SPIP et du JAP. Les directeurs de SPIP effectuent un travail remarquable qui n'est pas toujours apprécié à sa juste valeur. Il me paraît donc important de souligner, à l'occasion de l'examen de ce texte, les responsabilités éminentes qu'ils assument. Le troisième volet de la proposition de loi concerne les amendes forfaitaires, l'objectif étant d'en améliorer le taux de recouvrement. Le dispositif de l'amende forfaitaire a fait la preuve de son efficacité pour sanctionner des infractions « de masse », sans engorger les tribunaux. Il autorise une verbalisation immédiate et automatique de certaines infractions contraventionnelles, mais aussi de quelques infractions délictuelles, telles que la conduite sans permis ou sans assurance et l'usage illicite de stupéfiants. Afin d'accélérer leur recouvrement, la loi a prévu que le montant de l'amende forfaitaire due au titre de certaines infractions routières peut être minoré, si l'amende est réglée au moment de la constatation de l'infraction ou au plus tard dans un délai de quinze jours. Le contrevenant est ainsi incité financièrement à s'acquitter rapidement du montant de l'amende. Il est proposé d'élargir le mécanisme de l'amende forfaitaire minorée, en l'appliquant aux contraventions de la cinquième classe et en autorisant le pouvoir réglementaire à l'étendre à d'autres catégories de contraventions. Une autre disposition, plus ponctuelle, vise à éviter que les auteurs de certaines infractions routières échappent à une sanction, notamment à un retrait de points, parce que leur véhicule aurait été immatriculé, par erreur, sous le nom d'une personne morale. viens enfin au dernier volet du texte, qui s'inspire de suggestions formulées par la Cour de cassation dans son rapport annuel et qui présente un caractère assez technique. Il tend à simplifier le désistement de l'accusé ayant interjeté appel d'une décision de cour d'assises, à harmoniser le délai accordé au demandeur en cassation pour déposer un mémoire et à autoriser le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation à désigner le magistrat chargé de rapporter une affaire après le dépôt des mémoires des avocats, de manière qu'il soit plus facile de sélectionner le rapporteur le mieux à même de traiter le dossier. La commission a approuvé sans modification ces trois dispositions ponctuelles. Vous le voyez, mes chers collègues, ce texte cherche à parfaire des dispositifs existants qui sont déjà largement utilisés sur le terrain ou gagneraient à être développés. La commission des lois vous demande donc de l'approuver, tout en soulignant que d'autres mesures seront nécessaires pour faire vivre la promesse d'une justice de proximité : des mesures d'organisation, bien sûr, mais aussi l'allocation de moyens adaptés pour maintenir sur l'ensemble de notre territoire, notamment dans les territoires ruraux, des lieux de justice en nombre suffisant.

Aussi, toute évolution législative qui va dans le sens de son amélioration doit susciter notre attention et notre soutien. Les chiffres sont là, et ils ne sont pas bons ! Selon une étude de l'Institut français d'opinion publique (IFOP) réalisée en 2019, seul un Français sur deux déclare faire confiance à la justice, plaçant cette institution loin derrière les hôpitaux, l'armée, l'école ou la police. Plus problématique encore, 60 % des Français consultés dans la même étude considèrent que la justice fonctionne mal. Ces résultats nous interpellent toutes et tous, et nous préoccupent, car la justice est l'outil qui permet de réguler les conflits entre les individus et de pacifier les relations sociales. Elle contribue également, au quotidien, à garantir le respect de l'ordre républicain, des libertés publiques et des droits fondamentaux. Aussi, c'est avec un réel intérêt et de grandes attentes que nous avons accueilli cette proposition de loi relative à l'amélioration de la justice de proximité et de la réponse pénale.

alors que celles-ci ne représentent qu'environ 25 % du contentieux judiciaire en France. Nous regrettons donc que les affaires civiles et commerciales aient été écartées, lesquelles correspondent pourtant aux deux tiers des décisions de justice rendues chaque année.

Le second est la proximité temporelle, celle-là même qui permet de réduire le délai de traitement et d'audiencement des procédures en cours. C'est une période pendant laquelle un litige mineur peut devenir une source de contentieux majeur,

il faut des magistrats, il faut des greffiers, il faut du personnel administratif, il faut du personnel à la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). Or dans un classement réalisé par le Conseil de l'Europe sur les moyens alloués par habitant au budget de la justice, la France est classée au treizième rang des vingt-sept pays de l'Union européenne ce constat factuel nous montre les efforts substantiels qui restent à accomplir. Cela étant dit, nous vous donnons acte, monsieur le garde des sceaux, des crédits en hausse que vous avez obtenus dans le dernier projet de loi de finances ; nous formons le voeu que cette tendance haussière se confirme dans la durée.

Si je voulais être malicieux, j'y verrais un subterfuge visant à réduire artificiellement le stock d'affaires des JAP ... À côté de la

mais aussi réparer le préjudice. Elle doit réprimer justement l'auteur de l'infraction, veiller à la stricte application de la sanction prononcée et miser sur la capacité du condamné à se réinsérer dans la société, sans récidiver. C'est à cet idéal que nous souscrivons toutes et tous. L'ambition de cette proposition de loi est bien de tendre vers celui-ci, justement parce qu'elle vise à améliorer l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale. Mon expérience m'amène à témoigner de la complexité de nos dispositifs judiciaires, monsieur le garde des sceaux. Cette complexité met bien souvent en difficulté les victimes, en particulier celles qui ne sont pas accompagnées par un avocat ou une association. Pour nombre de ces victimes, chaque étape de la procédure, du dépôt de plainte jusqu'à la tenue du procès, relève du parcours du combattant et, lorsque ces procédures aboutissent, il n'est pas rare que la sanction et la réparation soient mises en oeuvre de façon aléatoire, renforçant un sentiment de défiance à l'égard de la justice.

Mais le manque de moyens ne saurait expliquer à lui seul les carences de la justice. Les mesures contenues dans notre code de procédure pénale sont perfectibles, et c'est bien à leur amélioration qu'a tenté de s'atteler cette proposition de loi. Ce texte, il est vrai, n'est pas révolutionnaire, il n'est pas non plus exempt de défauts- j'aurais l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Toutefois, il comporte plusieurs éléments bienvenus que notre collègue Alain Marc et vous-même, monsieur le garde des sceaux, avez soulignés. notamment de la mise en place à l'article 1 d'une possibilité de versement d'une contribution citoyenne à une association dédiée à l'aide aux victimes. La mise en valeur de ces structures associatives aura un double effet, puisqu'elles verront leur reconnaissance et leur place dans le paysage judiciaire renforcées.

Notre groupe est pleinement favorable à l'introduction à l'article 1 d'un stage de responsabilité parentale imposé par le procureur de la République aux personnes condamnées, parmi les peines édictées à l'article 41-2 du code de procédure pénale.

place centrale dans la procédure pénale. Malgré les réserves exprimées, nous avons souhaité, dans une démarche constructive, enrichir et compléter le texte. Notre vote dépendra en partie de l'accueil qui sera réservé à nos amendements.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, « Ouvrir une école, c'est fermer une prison » disait le grand poète Victor Hugo. S'il vivait en 2021, je suis sûr que le sénateur Victor Hugo préfèrerait cette formule : « ouvrir une prison, cela ne suffit plus, ouvrez-en plusieurs » ... À Amiens, Montpellier, Marseille ou Reims, dans toutes les villes et désormais les campagnes de France, les mêmes faits sont observés : des

La réforme que vous nous proposez aujourd'hui, monsieur le garde des sceaux, ne règle malheureusement pas le problème ! Certaines mesures vont certes dans le bon sens, comme la contribution financière demandée aux délinquants pour la réparation des dégâts qu'ils ont causés ou pour les associations de victimes, mais aussi une réponse pénale plus rapide pour les petites infractions. Mais comme d'habitude, vous n'allez pas au coeur et à la source du problème, puisque vous souhaitez faciliter et fluidifier le recours aux travaux d'intérêt général qui n'ont jamais empêché la récidive. On ne combat pas les barbares, en leur faisant balayer les rues,

aux travaux du pédopsychiatre Maurice Berger, qui explique qu'il faut traiter les primo-délinquants avec des peines d'enfermement dès la première condamnation. C'est la seule réponse qu'ils comprennent toutes les autres, et ils recommenceront ... Ils ne comprennent la loi que lorsqu'elle devient physique, quand elle les contraint, quand elle les punit, quand ils en ressentent sa force au quotidien. Même de courts séjours de quelques jours ou de quelques semaines peuvent éviter la récidive, y compris pour les plus jeunes. Près de la moitié des primo-délinquants ont entre treize et quinze ans : c'est à cet âge-là qu'il faut agir, qu'il faut sévir. La généralisation des TIG, c'est favoriser la récidive, pas la combattre ! Ce n'est pas l'enfermement qui engendre la récidive, mais bien les conditions

Cela pourrait être suffisant, si vous abandonniez votre xénophilie obsessionnelle, en expulsant les délinquants étrangers ! Il faut conclure. Incapable de tenir votre promesse et par conviction personnelle que l'enfermement doit être évité, vous souhaitez tout faire pour que les criminels évitent la prison. En attendant, ce sont les Français qui subiront votre laxisme dans les rues,

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, ces dernières années ; les nombreux faits divers nous le rappellent tous les jours. La montée de l'individualisme et le développement des incivilités du quotidien nuisent au vivre ensemble. Nous devons tous agir pour endiguer ce phénomène préoccupant les délais souvent trop longs de la réponse pénale, la permissivité de la société et l'incertitude de la peine n'ont rien arrangé. Les auteurs de cette proposition de loi ont cherché à apporter ont cherché à apporter une réponse concrète, rapide et certaine aux petits délits du quotidien. Je tiens à saluer cette volonté qui va dans le bon sens, car rien n'est pire que de donner un sentiment d'impunité à un primo-délinquant : c'est lui donner le permis de recommencer. Les mesures alternatives proposées dans ce texte sont fort intéressantes, en ce qu'elles proposent une réelle sanction et mettent l'auteur de l'infraction face à ses responsabilités. Dorénavant, ce dernier pourra, à la demande du procureur, réparer ses actes, en remettant en état les choses dégradées, en remettant l'objet du délit aux autorités, en n'entrant pas en relation avec la victime ou avec les complices ou encore en s'acquittant d'une contribution dite citoyenne.

Je me déplaçais très souvent sur les chantiers TIG de Tourcoing- rien de tel pour analyser l'impact des mesures réalisées ! -et les jeunes me présentaient quelques fois avec fierté leurs réalisations- travaux de peinture dans les écoles, rénovations de salles de sport, C'était souvent leur première expérience positive de vie, ils en étaient même surpris. Autrefois, seuls les petits boulots ingrats, voire dévalorisants, étaient proposés- c'était bien dommage.

La réussite de la mise en place de tels chantiers dépendait souvent de la confiance entre l'élu et le JAP. Il n'est pas toujours évident de trouver un interlocuteur et d'établir cette relation. J'espère donc que la simplification des règles relatives à l'exécution des TIG facilitera son déploiement.

individu sur deux ! Il est plus que temps de chercher des peines alternatives et de travailler collectivement. Il nous faut comprendre ce qui mène à la récidive et la façon La fonction essentielle de la sanction est d'acter la faute commise. La peine, quant à elle, permet d'intimider et de freiner les intentions néfastes. Les victimes doivent se sentir écoutées et, si celui qui leur a causé du tort est sanctionné, elles sont satisfaites. La prison reste incontournable dans certains cas, mais quoi qu'il en soit, sanctionner justement et rapidement demeure une obligation pour garantir l'avenir de notre pays.

La proximité permet de bien cerner son acte et sa prise en charge par une sanction adaptée. La police, si elle est organisée en proximité, donnera une analyse précise du contexte. Les magistrats et les avocats, s'ils sortent des universités locales, seront concernés par l'impact de leur travail autour du délinquant qu'ils connaissent bien. s'ils travaillent avec la PJJ et les élus locaux, la réaction sociale sera plus efficace. En revanche, la sanction doit rester ferme, forte, juste et surtout rapide.

Ainsi, dans son exposé des motifs est-il souligné la volonté de restaurer une justice de proximité luttant contre les incivilités et la délinquance quotidienne, en renforçant l'efficacité des réponses pénales. Cette ambition se matérialise notamment par l'ajout de nouvelles mesures alternatives aux poursuites et par la simplification des règles concernant la mise en oeuvre des travaux d'intérêt général. L'article 1, par exemple, qui insère des mesures de réparation accomplies en faveur de la victime, est une belle initiative.

auprès d'une association d'aide aux victimes et il prévoit la mise en place de mesures de réparation, de restitution ou de remise en état des lieux ou des choses dégradées. dégradées. Cela permettra de faciliter l'indemnisation des collectivités territoriales qui doivent en supporter les coûts. notre bord politique dans cette assemblée, nous ne pouvons que nous associer à cette initiative. En effet, si l'ensemble des mesures alternatives aux poursuites représente 40 % à 50 % des réponses pénales en France, elles permettent une solution pénale rapide qui a tout son intérêt face au manque d'efficacité souvent décrié de notre système pénal. En outre, nous estimons que les mesures de réparation et de TIG devraient être préférées à celles privatives de liberté, en ce qu'elles permettent de lutter contre la politique du « tout carcéral

L'article 1 , adopté en commission à l'Assemblée nationale, élève à cent heures le plafond des heures de travail non rémunéré pour les TIG.

Ces deux dispositions constituent un recul sur les droits de la personne condamnée que nous ne pouvons pas accepter. De surcroît, les alinéas 3 et 4 de l'article 2

Nous regrettons, une fois encore, que sans moyens humains et matériels conséquents, notre justice ne soit pas en capacité d'améliorer la qualité de sa réponse pénale. Si ce texte relève d'une bonne intention, celle-ci reste toutefois privée des outils nécessaires à sa réussite. Nous nous opposons également aux dispositions dont j'ai déjà fait état. Mes chers collègues, le rendez-vous avec la modernisation de notre justice

Elle vise cette petite délinquance qui, des incivilités aux délits de faible gravité, peut véritablement gâcher la vie de nos concitoyens. Cette délinquance doit être traitée avec rapidité et efficacité, d'abord parce qu'une réponse judiciaire tardive entraîne bien souvent une désaffection à l'égard de la justice d'une partie de la population, victime ou témoin de cette délinquance du quotidien, voire son ressentiment ensuite parce qu'il est indéniable que la vertu pédagogique d'une sanction s'évanouit à mesure que celle-ci s'éloigne de la date de commission des faits. le présent texte procède-t-il à plusieurs ajustements visant principalement à compléter les mesures alternatives aux poursuites et les mesures de composition pénale. Il met en place des outils tels que la remise en état ou le versement d'une contribution citoyenne à une association agréée d'aide aux victimes. Il simplifie le régime du travail d'intérêt général afin de favoriser le recours à ce type de peine et de réduire son délai d'exécution en confiant cette mission aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP). Il est important de rappeler que le juge d'application des peines pourra toujours décider de conserver sa compétence. La proposition de loi améliore également la procédure de l'amende forfaitaire afin d'accélérer son recouvrement, en intégrant, dans le champ de la minoration de son montant, l'ensemble des contraventions prévues par le pouvoir réglementaire. Enfin, en compte des observations formulées par la Cour de cassation depuis 2017, le texte simplifie la procédure applicable en appel et en cassation. La commission des lois du Sénat a procédé à quelques précisions. À cet égard, nous nous félicitons qu'elle ait retenu l'amendement de notre groupe visant à permettre à l'État de mettre à disposition des associations, des fondations reconnues d'utilité publique ou des organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement des biens immeubles dont il est devenu propriétaire dans le cadre d'une procédure pénale. Cet amendement s'inspirait d'une disposition déjà approuvée lors de l'examen de la proposition de loi

Nous vous proposerons deux autres amendements, que nous aimerions également voir adopter. Le premier tend à prévoir que, dans le cadre d'une mesure alternative aux poursuites, l'auteur des faits de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit au bénéfice d'une personne morale à but non lucratif désignée par le procureur de la République.

Il est vrai que les dispositions contenues dans cette proposition de loi n'entraîneront pas une révolution de la justice pénale, de l'aveu même de l'auteur du texte, mais elles auront, j'en suis convaincu, une grande utilité éducative et pédagogique, ce qui permet bien souvent de prévenir la récidive et encourage la réinsertion. Cette proposition de loi s'inscrit en outre, comme l'a souligné le rapporteur, dans la dans la droite ligne de l'engagement politique majeur pris par le Premier ministre lors de son discours de politique générale, le 15 juillet 2020. Des moyens accompagnent cette volonté politique, puisqu'un budget de 200 millions d'euros a été spécialement alloué à cet effet dans le projet de loi de finances pour 2021.

Vous y préconisez le recours aux audiences foraines lorsque le flux d'affaires le justifie ou encore un approfondissement des relations avec les partenaires locaux. En conclusion, cette proposition de loi est non seulement le fruit d'un travail avec les acteurs judiciaires et pénitentiaires, mais également un exemple de coconstruction législative entre le Parlement et le Gouvernement,

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, une fois de plus, ce texte illustre la façon dont le Gouvernement continue de légiférer en matière de justice dans un calendrier législatif restreint, comme en témoigne la parfaite cohérence, monsieur le garde des sceaux, entre la présente proposition de loi et votre circulaire de politique pénale en date du 15 décembre dernier.

pour effectuer un travail de qualité et réduire la surcharge. Deuxièmement, les procureurs ne sont toujours pas indépendants, la réforme de l'indépendance du parquet n'ayant toujours pas été engagée. Il nous paraît important d'avancer concrètement en matière d'indépendance du procureur de la République : s'il se voit attribuer plus de compétences, il se doit d'autant plus d'être neutre dans son essence et impartial dans ses décisions.

à mettre à disposition de certaines associations ou fondations d'utilité publique ou à des organismes qui concourent à la politique du logement des biens immobiliers saisis ou confisqués dans le cadre d'une procédure pénale. Nous considérons que ces mesures sont plutôt positives et qu'elles améliorent le texte. En outre, nous partageons pleinement la conclusion du rapporteur Alain Marc sur le texte : « Les mesures envisagées par la proposition de loi ne suffiront pas à concrétiser la promesse d'une justice de proximité : rapprocher la justice du justiciable passera davantage par des mesures d'organisation, par le maintien des lieux de justice au plus près des territoires et par l'allocation de moyens adaptés qui permettront de réduire les délais de jugement et d'apporter une réponse à chaque infraction.

qu'est avancée de façon récurrente la nécessaire célérité de la justice, que l'excessive durée du procès pénal ne peut pas être le seul et unique argument pour donner davantage de pouvoirs aux procureurs. Pour l'ensemble de ces raisons, nous nous abstiendrons sur ce texte.

La proximité est une manière d'être, un comportement, mais n'est pas en elle-même un programme d'action. J'avoue lui préférer depuis bien longtemps, dans nos gestions locales, la notion d'« accessibilité », tout simplement, et, en matière de justice, de respect du justiciable, comme de tout usager. En d'autres termes, la justice doit être accessible ; je ne suis pas sûr, monsieur le garde des sceaux, qu'elle doive être proche. J'en viens à l'esprit du texte et et à son contenu. Vous proposez de perfectionner la panoplie des alternatives aux poursuites, c'est bien sûr une bonne chose. Vous proposez également une contribution citoyenne.

Je ne veux pas dire par là que nous assistons à un début d'américanisation de notre système judiciaire. Je vous donne volontiers acte, monsieur le garde des sceaux, qu'avec une limite à 3 000 euros, nous sommes très loin d'une telle situation.

Nous savons tous que ce qui relève du droit de la peine est par essence de nature législative. Il est donc normal que l'ensemble de ces éléments soient soumis au Parlement.

des autorités administratives indépendantes, des agences, c'est-à-dire de toutes les formes de démembrement de l'État. Une vieille règle très connue dans les collectivités locales, qui vaut également à l'échelle de l'État, veut qu'une institution, une fois créée,

qu'il aura fallu ce texte pour me permettre d'appréhender la différence de nature juridique entre les travaux d'intérêt général et les travaux non rémunérés. Cette subtilité ne m'avait pas frappé

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, en fin d'année dernière, plus de la moitié de nos concitoyens déclaraient dans un sondage ne pas avoir confiance en la justice. Ils sont en effet nombreux à décrier sa lenteur et à exprimer le ressenti d'un manque d'efficacité. Cette situation est préoccupante en elle-même, en elle-même, d'autant plus que la justice constitue, vous le savez tous, mes chers collègues, l'un des fondements les plus essentiels de l'État de droit. Quand elle fonctionne mal, c'est tout l'édifice qui est fragilisé. La confiance que les citoyens placent dans l'appareil judiciaire, mais aussi dans le politique et dans les élus, s'érode. Il est impératif de remédier à cette situation, qui ne date malheureusement pas d'hier. Elle est notamment due à un manque chronique de moyens. Le Gouvernement a commencé à y répondre en augmentant significativement le budget destiné à la justice en 2021. Cet effort, que nous saluons, devra se poursuivre dans la durée pour que la justice de notre pays retrouve une pleine efficacité. En plus d'un indispensable effort budgétaire, il faut également simplifier notre droit et rapprocher la justice des citoyens.

Mineures par leur degré, elles posent cependant un problème majeur, tout d'abord par leur nombre, car elles représentent près de la moitié de l'activité des parquets, majeur, ensuite, du fait de l'importance que revêt le traitement de ces infractions du quotidien. Ces dernières empoisonnent la vie de nos concitoyens. En l'absence de réponse judiciaire rapide, elles laissent prospérer dans les territoires un sentiment d'impunité délétère, tant pour ceux qui commettent ces infractions que pour ceux qui les subissent. « Faire une loi et ne pas la faire exécuter, c'est autoriser la chose qu'on veut défendre », disait Richelieu. Ces petites infractions doivent donc recevoir une réponse rapide et adaptée si nous voulons accroître le respect de la loi. Le texte que nous examinons comporte à cet égard des améliorations bienvenues. L'élargissement proposé des alternatives aux poursuites pénales prend en considération les intérêts de la victime, que ce soit par la réparation de son préjudice ou par la contribution de l'auteur de l'infraction Ces dispositifs responsabilisent l'intéressé et favorisent également son insertion et son amendement. Ces petites infractions constituent parfois de premiers pas vers la délinquance. Y répondre avec réactivité et pédagogie permet sans nul doute de réduire les risques de réitération. Outre ces nouvelles mesures, le texte prévoit des simplifications de procédures existantes dans l'objectif de raccourcir les délais. La composition pénale pour les infractions contraventionnelles ne devra plus être validée par un magistrat du siège,

Afin d'améliorer le recouvrement des amendes, le texte prévoit en outre de minorer le montant des amendes des contraventions de cinquième classe lorsque l'intéressé s'en acquitte dans les délais. La majoration, comme la minoration, incite les personnes concernées à régulariser leur situation. La commission des lois a enrichi le texte avec d'utiles dispositions. À cet égard, nous saluons l'excellent travail de notre rapporteur, Alain Marc. Les dispositions contenues dans ce texte amélioreront l'efficacité de notre justice pénale. Aussi notre groupe soutiendra-t-il leur adoption.

Par ailleurs, demander à l'auteur des faits de ne pas rencontrer les coauteurs ou complices est une interdiction de toute évidence impossible à faire respecter, même si l'intention est très louable. En effet, on imagine mal les procureurs mobiliser pour ce faire des gendarmes, qui ont autre chose à faire. Cette mesure décrédibilise une fois de plus l'action de la justice, qui n'en a pas besoin. Ensuite, demander à l'auteur des faits de s'acquitter d'une contribution citoyenne auprès d'une association d'aide aux victimes peut paraître gênant. Comment choisir cette association sans entrer dans des considérations subjectives ? Selon quels critères ?

spécialisations et, aujourd'hui, marche arrière vers une justice de proximité, civile, pénale, géographique, plus rapide : les auxiliaires de justice sont épuisés par cette nouvelle réalité qui dévore toute leur énergie. À peine ont-ils mis en oeuvre une loi qu'une autre intervient

comme bon nombre de sénateurs, je voue une admiration sans bornes à celui qui fut et reste le plus grand d'entre nous : je veux parler du sénateur Victor Hugo. Au début de cette discussion générale, notre collègue Ravier ayant cru bon, de façon hasardeuse, de le faire parler plus d'un siècle après

Mais revenons-en à notre proposition de loi. Dans nombre de nos territoires, la délinquance, les incivilités, l'insulte, le petit trafic, les troubles à ce que le code communal appelle la « tranquillité publique » se sont développés au point de gâcher la vie de nos concitoyens. Faute d'une réponse judiciaire, une forme d'impunité s'est peu à peu installée, entraînant automatiquement une croissance exponentielle de ces méfaits. Trop souvent, bien trop souvent, les victimes ont le sentiment que ces actes de délinquance restent impunis. Trop souvent, nos forces de l'ordre ont l'impression de courir toujours après les mêmes individus. Trop souvent, enfin, les délinquants ont un sentiment d'impunité quasi totale face à ceux qui Nous rappelons régulièrement dans cet hémicycle la réalité de cette délinquance du quotidien qui reste sans réponse. Selon le sondage de l'IFOP de septembre 2020, plus de 73 % des Français interrogés estiment que la justice n'est globalement pas assez sévère. sévère. Oui, cette proposition de loi est bienvenue s'il s'agit d'apporter une réponse judiciaire rapide et en proximité. l'instauration de mesures alternatives visant à rendre la justice plus efficace pour répondre dans des délais rapides à certaines de ces infractions en évitant un procès est une ambition que nous partageons. faciliter le recours à la peine de travail d'intérêt général s'inscrit dans cette logique. Aux actes commis, il faut apporter une réponse rapide et systématique. Une justice plus proche de leur quotidien au coeur des territoires, des villes et des quartiers : voilà ce que nous demandent les Français. Ce traitement en temps réel, conçu comme un instrument de maîtrise de l'action publique au service des parquets permettrait par ailleurs d'accélérer le cours de la justice pénale. Notre justice sera d'autant plus efficace que les délais entre la commission de l'infraction et la réponse judiciaire seront brefs, mais cette conception globale et moderne de l'action publique suppose une adaptation de l'organisation des parquets à la procédure de traitement en temps réel et, bien entendu, l'affectation de nouveaux moyens. Elle impose également que les relations partenariales avec les collectivités locales, le tissu associatif et les acteurs de terrain soient renforcées, comme vous l'avez rappelé, monsieur le garde des sceaux. Le projet de création d'une contribution citoyenne plafonnée à 3 000 euros au bénéfice d'une association d'aide aux victimes est une proposition qui va également dans le bon sens. Celui qui commet une infraction doit en payer le prix dans tous les sens du terme,

Allons-nous enfin nous donner les moyens de réagir face au désordre qui s'installe insidieusement et fait le lit des extrêmes ? Une partie de la réponse est aujourd'hui dans entre nos mains, mes chers collègues ; l'autre dépendra du courage et de la volonté du Gouvernement et des juges de faire appliquer ces nouvelles dispositions.

L'attente de la population est forte. Cette proposition de loi pourrait y apporter quelques premiers éléments de réponse. En cherchant à améliorer l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale, elle prévoit de « muscler » les peines alternatives pour nous assurer de l'efficacité de leur prononcé. Dans son ensemble, ce texte propose des ajustements évidemment souhaitables. Il faut indéniablement renforcer la justice dans sa proximité et sa rapidité. Cette proximité trouve une forme innovante au travers de la mise en place d'une contribution citoyenne versée par l'auteur des faits en faveur d'une association d'aide aux victimes. Cette nouvelle disposition est la bienvenue, car elle sera un bon moyen de sensibiliser les auteurs d'infraction, notamment les plus jeunes, qui ne prennent pas toujours la mesure de leurs actes. L'élargissement des possibilités laissées au procureur en matière de composition pénale mérite aussi un accueil favorable. Cela vaut pour l'augmentation du plafond des heures de travail non rémunéré autant que pour l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale. De même, s'agissant de la procédure pénale, mes collègues du groupe du RDSE et moi-même accueillons favorablement les différentes mesures proposées, qu'il s'agisse de l'extension du dispositif de minoration des amendes forfaitaires, de la constatation du désistement d'appel en matière criminelle ou encore de la désignation des conseillers rapporteurs de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Sans doute ne suis-je pas assez spécialiste pour me prononcer sur l'opportunité technique de toutes ces mesures, mais il y a lieu de penser qu'elles seront bienvenues, les travaux de notre rapporteur l'ont mis en évidence. au-delà de son intérêt pratique pour les services judiciaires ou pénitentiaires, ce texte m'a inspiré deux réflexions plus générales. En premier lieu, cette proposition de loi s'inscrit dans une tendance profonde, à savoir le renforcement les mesures alternatives. Ainsi, la place du procès recule, comme celle du juge. À force de petites touches éparpillées, le tableau de notre justice pénale se transforme sensiblement. Cette multiplication des textes en faveur des mesures alternatives doit nous conduire à nous interroger sur la place du procès pénal dans notre cité. À trop renforcer l'alternative, nous ne devons pas en oublier le principal : une composition pénale n'est pas un jugement, et le bureau d'un procureur ne s'apparente pas à une salle d'audience. Tout cela participe d'une forme de « déritualisation » du règlement des suites de l'infraction. Il ne faudrait pas que l'éviction des formes traditionnelles conduise, à terme, à l'exclusion de tout formalisme.

si elle n'est pas accompagnée d'une volonté politique sérieuse et d'envergure, et donc de moyens humains et matériels. La délinquance quotidienne n'est pas une affaire de légistique, d'organisation des compétences ou de panel des sanctions. Répondre à la délinquance, c'est également répondre à la précarité, à la marginalisation, à la souffrance sociale. Cette délinquance du quotidien est aussi un appel à l'éducation. Tels sont les axes auxquels nous devons consacrer du temps pour nourrir efficacement l'espoir que la tendance s'inverse.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

est à Mme Esther Benbassa. Le présent amendement est inspiré d'une initiative locale, que je salue, et qui gagnerait à se développer et à se généraliser à tout le territoire. En effet, l'intégration d'un stage spécifique de sensibilisation à la protection de l'environnement dans la liste des stages susceptibles d'être mis en oeuvre sur le fondement de l'article 41-1 du code de procédure pénale me tient tout particulièrement à coeur en tant qu'écologiste. En Savoie, par exemple, le parquet de Chambéry organise depuis déjà plus d'un an, au bord du lac d'Aiguebelette, des stages de citoyenneté environnementale pour les pour les auteurs d'infractions commises dans des milieux naturels. Ainsi, dix hommes et deux femmes d'âge et d'origine sociale divers ont pu bénéficier de cette expérience de sensibilisation aux problématiques environnementales locales. Cette initiative a également été reprise en Charente-Maritime.

aux personnes morales à but non lucratif le bénéfice du dessaisissement de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit. Plusieurs garanties sont prévues afin de ne pas créer d'insécurité juridique : d'une part, la personne morale sera désignée par le procureur de la République et, d'autre part, la chose dessaisie à son bénéfice ne pourra être qu'une chose dont l'auteur des faits est propriétaire et sur laquelle aucun tiers n'est susceptible d'avoir des droits.

ou qui en est le produit. Nos collègues du groupe RDPI proposent que le bien ayant fait l'objet d'une telle mesure de dessaisissement puisse être attribué à une personne morale à but non lucratif désignée par le procureur de la République, à condition que le bien appartienne à l'auteur de l'infraction afin d'éviter toute difficulté en cas de demande de restitution formulée par la victime de l'infraction.

d'une reconduction de ce délai de six mois paraît beaucoup trop lourd. Pour des faits plus graves qui nécessitent une protection renforcée de la victime, il convient de saisir le tribunal correctionnel qui pourra prononcer une interdiction pour une durée plus longue. Un contrôle judiciaire peut également prévoir une interdiction de contact. Enfin, dans un contexte de violences conjugales, le juge aux affaires familiales peut également délivrer une ordonnance de protection prévoyant une telle mesure. Ainsi, certaines procédures qui existent déjà permettent d'atteindre l'objectif que vous visez.

Cet amendement tend à affilier à la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale les personnes qui effectuent un travail non rémunéré dans le cadre d'une transaction conclue avec le maire, comme le permet l'article 44-1 du code de procédure pénale. Si le code de la sécurité sociale prévoit l'affiliation des condamnés effectuant un TIG ainsi que celle des personnes effectuant un TNR dans le cadre d'une composition pénale, il ne vise pas l'hypothèse de la transaction avec le maire, ce qui oblige les communes qui ont recours à cette mesure à souscrire une assurance privée pour couvrir les éventuels frais de santé qui seraient occasionnés par un accident ou un problème de santé survenu à l'occasion du travail. Cet amendement vise à réparer cette omission, afin d'inciter les communes à utiliser ce dispositif qui présente un intérêt pour prévenir la récidive et favoriser la réinsertion sociale et professionnelle des personnes concernées. Quel est l'avis du Gouvernement ? Comme je l'ai

2021. Sont visées les compositions pénales qui peuvent être proposées à des mineurs délinquants sous réserve de certaines adaptations de procédure. Le code de procédure pénale est modifié afin d'ajouter le stage de responsabilité parentale à la liste des stages pouvant être effectués dans le cadre d'une composition pénale. Ce stage peut présenter un intérêt pour de très jeunes parents qui rencontreraient des difficultés pour assumer de façon satisfaisante leurs responsabilités éducatives. Il est donc logique de le faire figurer également dans le code de la justice pénale des mineurs. Plutôt que d'allonger la liste des stages visés par ledit code, l'amendement tend à introduire une rédaction plus synthétique, ce qui évitera d'y revenir si d'autres stages sont ajoutés par la suite. La deuxième modification est purement formelle et tire les conséquences de l'ajout d'un alinéa à l'article 41-2 du code de procédure pénale.

En effet, ces dispositions ont pour objet de transférer la compétence en matière de détermination des modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, jusqu'alors détenue par le juge de l'application des peines,

un travail d'intérêt général doit se soumettre à un examen médical préalable, dans le but de rechercher si elle n'est pas atteinte d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s'assurer qu'elle est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de l'affecter. Cet examen médical constitue une protection du condamné, puisqu'il permet de s'assurer que la personne est médicalement apte au travail, notamment pour des activités physiques qui peuvent parfois être pénibles. Rappelons par exemple que le travail d'intérêt général est une peine qui peut être proposée à l'auteur de certaines infractions ayant au moins 16 ans au moment du jugement. De fait, de jeunes personnes peuvent être concernées par une telle peine, mais il peut aussi s'agir de personnes ayant atteint un âge où certaines tâches sont susceptibles de s'avérer difficiles à effectuer. Or, par les dispositions du présent article, il est proposé de supprimer le caractère systématique de l'examen médical sous prétexte de simplifier la mise en oeuvre des TIG. Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 5 du présent article,

qui prévoit que la procédure d'affectation d'un condamné sur un poste de travail d'intérêt général relève de la compétence du directeur du SPIP, sauf si le juge de l'application des peines décide d'exercer cette compétence. Par cohérence, cet amendement a pour objet de prévoir à l'article 2 que, en cas de compétence du directeur du SPIP, l'établissement de la liste des postes de TIG ne relève pas du JAP, mais bien du directeur du SPIP. Celui-ci dispose en effet d'une équipe étoffée

comme le prévoit explicitement l'article.

Quant à l'amendement n° 15, le texte adopté par la commission prévoit que le directeur du SPIP est compétent pour instruire les demandes des employeurs qui souhaitent proposer des TIG, et pour établir la liste de ceux qui sont offerts dans le département, sauf si le juge de l'application des peines décide de statuer lui-même sur une demande. L'amendement de nos collègues objet de supprimer cette possibilité d'intervention du juge de l'application des peines. On continuerait de consulter le JAP, mais c'est au directeur du SPIP, et à lui seul, que reviendrait la décision de trancher sur la demande qui lui est soumise.

Dans son quatrième alinéa, l'article 10-2 du code de procédure pénale prévoit qu'une victime qui vient déposer plainte doit être informée de son droit d'être assistée par une association ; et dans son huitième alinéa, qu'elle peut être accompagnée à tous les actes de la procédure par une personne de son choix.

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'élection du président de la République 354). J'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de ce texte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

jamais votre assemblée n'aura, dans son histoire récente, examiné en aussi peu de temps autant de textes électoraux : la loi organique du 24 décembre 2020 relative aux délais d'organisation des élections législatives et sénatoriales partielles, loi portant report du renouvellement général des conseils départementaux et des conseils régionaux que vous venez d'adopter définitivement et, cet après-midi, le projet de loi organique relatif à l'élection du président de la République. Les deux textes de report devaient gérer l'immédiat, l'urgence de concilier impératifs démocratiques et impératifs sanitaires. Vous les avez examinés dans un esprit foncièrement républicain, dans un esprit de rassemblement et de responsabilité, au moment où notre pays reste confronté à une crise sanitaire sans précédent. Le projet de loi organique que vous examinez ce soir nous invite, pour sa part, à renouer avec une forme de « normalité démocratique » tout en nous projetant résolument dans l'avenir. le texte procède, comme chaque année qui précède l'élection présidentielle, à l'actualisation de la loi organique du 6 novembre 1962, afin de rendre applicables au scrutin présidentiel les évolutions des règles du code électoral, intervenues depuis la dernière élection. Il permet aussi, comme chaque fois, de tenir compte des remarques formulées par le Conseil constitutionnel à l'occasion du dernier scrutin. Ces adaptations ont été examinées par votre commission des lois et ne posent pas de problème de principe, puisqu'elles s'en tiennent, pour l'essentiel, à l'application du droit commun. Ce souhait de s'en tenir au droit commun explique que le Gouvernement ait défendu, par exemple, au cours de l'examen parlementaire de ce texte, le fait d'écarter le recours à la double procuration. Il

Je sais que cette préoccupation est largement partagée par votre assemblée et nous aurons l'occasion d'y revenir, lorsque nous examinerons l'amendement de M. Mouiller.

Au-delà de ces innovations, les discussions parlementaires qui se sont tenues à l'occasion de l'examen des différents projets de loi ont confirmé l'intérêt porté par toutes les formations politiques à la question des nouvelles modalités de vote.

le Gouvernement a cherché à proposer une troisième voie qui concilie l'ensemble des contraintes, grâce à un dispositif qui simplifie et renforce la participation tout en assurant un vote personnel et secret, respectueux de la sincérité globale du scrutin.

d'abord, il porte sur une élection, certes structurante, mais qui reste extrêmement simple dans son principe : quelques candidats sont départagés dans une circonscription unique par l'ensemble des électeurs.

Ensuite il s'agit d'une élection qui mobilise, et pour laquelle les Français seront heureux que les modalités de vote soient facilitées, afin de leur permettre d'y participer le plus largement possible. Le dispositif que nous proposons vise, comme vous le savez, à offrir la possibilité aux électeurs et aux électrices qui le souhaitent de voter sur une machine électronique, quelques jours avant le scrutin présidentiel. Ce dispositif, très innovant,-

afin d'adapter les règles de cette élection majeure aux évolutions de notre droit électoral, pour sécuriser la campagne électorale et les opérations de vote, sans pour autant

Elle a ainsi adopté le renvoi à un décret simple, en lieu et place d'un décret en conseil de ministres, de la convocation des électeurs, afin de préserver l'esprit de l'article 7 de la Constitution. La commission a également créé une obligation pour les instituts de sondage de publier leurs marges d'erreur. Un autre point saillant de nos discussions

à l'élection du président de la République. Aussi, afin d'éviter un certain nombre de difficultés sur la ventilation entre les dépenses engagées par un éventuel même candidat aux élections régionales, départementales la commission a proposé, par sagesse, de ramener au 1 juillet 2021 le début de la période de financement de l'élection présidentielle. Madame la ministre, j'avais prévu d'entrer dans le détail de ces avancées techniques. Malheureusement, un événement est venu contrarier ce projet.

En second lieu, l'amendement que vous proposez souffre d'incomplétude, laissant beaucoup de questions en suspens. Quel serait le nombre de machines à voter disponibles afin d'assurer un maillage territorial satisfaisant ?

Par définition, un vote par anticipation signifie que la campagne officielle ne sera pas terminée au moment où certains électeurs accompliront leur devoir civique. Or, si un événement marquant venait à bouleverser au dernier instant la formation du jugement de l'électeur- je pense notamment au débat entre les deux tours -, ce dernier ne pourra pas revenir sur son vote. Ainsi, plus la période d'anticipation sera importante, plus le risque du changement d'opinion sera élevé. D'autant que la formation du jugement des électeurs peut intervenir très tardivement dans dans le cadre du processus électoral, parfois même dans les dernières heures. Malheureusement, ce vote par anticipation ne tient pas compte de cette réalité. D'un point de vue constitutionnel, j'aimerais ajouter que le fait que les électeurs ne disposent pas des mêmes éléments d'information, le jour de l'élection, entraîne inévitablement une rupture d'égalité entre eux qui eux qui peut porter atteinte à la sincérité du scrutin, et donc à la légitimité du candidat élu. Cela est d'autant plus vrai lorsque l'écart de voix entre les deux candidats est minime. Par définition, le vote par procuration est diffus, car les électeurs ne sont pas confrontés au même instant électoral, ce qui me conduit à penser que cette disposition peut être très fragile constitutionnellement.

Le Conseil constitutionnel, juge de l'élection présidentielle avait d'ailleurs souligné, dans l'une de ses décisions, que l'usage de ces machines à voter soulevait un réel problème de fiabilité, lié notamment à l'impossibilité

de plus en plus vieillissant, mais qui se refusent à investir sans avoir la certitude de la pérennisation du système. J'ajoute que l'absence que l'absence de bulletins de vote papier empêche tout recomptage. Il faudra donc faire confiance aux informaticiens pour s'assurer de l'absence d'un quelconque piratage. On peut enfin émettre des doutes sur le déroulement du dépouillement le jour même du scrutin : cela implique en effet que les machines à voter seront stockées dans les mairies pendant plusieurs jours avec le résultat des votes en mémoire, ce qui peut ouvrir la porte à des fraudes. porte à des fraudes. Je dirai un dernier mot, enfin, sur les effets sociologiques de cet amendement. On peut se demander légitimement si cette procédure ne favorise pas le vote des électeurs urbains appartenant à une catégorie socioprofessionnelle supérieure, ceux-là mêmes qui pourront se permettre de prendre une demi-journée de RTT en pleine semaine pour se rendre dans l'un des rares bureaux de vote du territoire, avant tout simplement de partir en villégiature le week-end. Même si nous devons nous interroger sur l'évolution des modalités des opérations de vote, il est certain que cela ne saurait être la seule réponse à l'abstention grandissante : est-ce le mode d'organisation du scrutin qui crée l'abstention ? Non, incontestablement non ! Je pense que le désamour de nos concitoyens à l'égard de la politique est beaucoup plus profond.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, ce projet de loi nous donne l'occasion de débattre des conditions de la tenue de la prochaine élection présidentielle un an à peine avant le scrutin. Nous sommes nombreux, élus locaux et électeurs, à nous inquiéter des orientations prises par le Gouvernement.

La sincérité du scrutin dépend aussi de la sincérité et de l'égalité entre les candidats durant la campagne : la partie est donc plutôt mal engagée. À toutes fins utiles, je rappelle que les conseillers départementaux et régionaux peuvent, comme les maires et les parlementaires, parrainer un ou une candidate à l'élection présidentielle. Les élus locaux conditionnent la campagne présidentielle, ne l'oublions pas ! Les débats qui ont eu lieu sur ce texte pour faire évoluer le code électoral vers la double procuration, le vote électronique, le vote par correspondance, ou encore le vote par anticipation, ne constituent pas un renforcement, mais un affaiblissement de la démocratie. Le déplacement dans les bureaux de vote doit être privilégié, car l'électeur doit rester un acteur vivant de la vie démocratique. Voter est un droit, mais aussi un devoir civique La première condition pour que les citoyens retrouvent le chemin des bureaux de vote est la confiance, notamment dans la fiabilité de l'organisation des scrutins, dans celle du scrutin présidentiel. L'image désastreuse laissée par les soupçons de fraude lors de l'élection présidentielle américaine, à cause du vote par correspondance, doit nous conduire à rejeter cette option : il faut pour protéger la sincérité du scrutin et préserver la confiance des électeurs. L'expérimentation du vote électronique, très minoritaire et très contesté, loin d'être étendue, doit également prendre fin dans notre pays. Le Royaume pays de naissance des « machines à voter », a lui-même fini par interdire ce procédé en raison de la fraude qu'il pouvait susciter. Par ailleurs, l'établissement de procurations donne déjà lieu à de nombreuses situations très critiquables. L'affaire dite des « fausses procurations dans les Ehpad », qui met en accusation élus, candidats et militants de la droite dite

La crise sanitaire a été l'occasion pour le Gouvernement de confisquer un certain nombre de nos libertés économiques, individuelles et démocratiques. L'épidémie ne doit pas justifier une nouvelle attaque en règle contre la démocratie en bradant notre droit électoral.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, chaque élection présidentielle sous la VRépublique a marqué notre histoire républicaine. Cela s'explique par le rôle joué par le Président de la République, qualifié par Michel Debré de « clé de voûte » de nos institutions, et par l'organisation, à compter de 1965, d'un scrutin au suffrage universel garantissant un lien direct entre les électeurs et le chef de l'État. L'importance de cette élection se traduit par le niveau des normes qui en arrêtent les modalités. Les principales règles relatives à l'élection présidentielle sont fixées par l'article 7 de la Constitution, ainsi que par la loi organique du 6 novembre 1962. Les règles de l'élection présidentielle doivent s'adapter aux évolutions de notre droit électoral depuis son adoption par référendum, la loi du 6 novembre 1962 a déjà été modifiée à vingt-trois reprises. Depuis 1988, chaque élection présidentielle est précédée d'une adaptation législative. usage est ancré dans notre tradition républicaine, notamment pour prendre en compte les observations du Conseil constitutionnel sur la précédente

Le projet de loi organique qui nous est présenté, comme le veut l'usage plus d'un an avant le scrutin, constitue ainsi un texte de réglage qui comporte divers ajustements ajustements techniques dans la perspective de l'élection présidentielle du printemps 2022. Il comprend plusieurs axes. L'article 1 concerne les opérations préparatoires au scrutin. Il fixe notamment le délai de convocation des électeurs à dix semaines avant le premier tour de l'élection. L'article 2 reporte en outre à 2027 la procédure dématérialisée de transmission des parrainages annoncée en 2016, en raison du retard pris dans l'identification numérique des citoyens. Il s'attache également aux règles de financement de la campagne et prévoit la dématérialisation des « reçus-dons » et du dépôt des comptes de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Enfin, cet article concerne le vote par correspondance des détenus, qui peuvent aussi bénéficier d'une autorisation de sortie pour voter ou établir une procuration.

Sous la responsabilité de qui seront-elles placées ? Qui les paiera ? Avons-nous le même avis une semaine avant le vote et le jour même du scrutin ? Pourquoi le Gouvernement n'a-t-il pas fait état de ce nouvel amendement lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines ? Par ailleurs, les articles 2 et 3 procèdent à plusieurs actualisations à la suite d'évolutions intervenues dans le code électoral : l'inscription sur les listes électorales sera possible jusqu'au sixième vendredi avant le scrutin ; le droit de vote est maintenu pour les majeurs sous tutelle ou curatelle ; les dons sur les plateformes numériques seront autorisés. On notera une modification importante : la « déterritorialisation » des procurations rendue possible par la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. Enfin, un dernier volet du texte a trait à l'inscription sur les listes électorales consulaires. Je me félicite que notre commission des lois ait apporté un certain nombre de modifications qui sont venues enrichir ce texte. Je suis heureux notamment qu'elle ait souhaité éviter tout chevauchement avec les comptes de campagne des élections régionales et départementales de juin 2021, en faisant débuter la période de financement de l'élection présidentielle au 1juillet 2021. Je me réjouis également qu'elle impose aux instituts de sondage de publier leurs marges d'erreur et qu'elle confère un caractère expérimental à la dématérialisation des comptes de campagne de l'élection présidentielle. J'approuve aussi la commission lorsqu'elle souhaite que les électeurs soient convoqués par décret simple plutôt que par décret en conseil des ministres, par cohérence avec l'article 7 de la Constitution. Enfin, je la rejoins lorsqu'elle entend permettre aux présidents des conseils consulaires des Français de l'étranger et des conseils exécutifs de Corse et de Martinique de parrainer un candidat à l'élection présidentielle, et lorsqu'elle rend obligatoire

voici donc une loi organisant l'événement qui est dans l'esprit de tous, mais de certains plus que d'autres, comme l'ont montré les récentes manoeuvres au sein de notre hémicycle : l'organisation de la prochaine élection présidentielle. Ce texte prévoit la convocation par décret de cette élection dix semaines avant le premier tour, date de départ du dépôt des parrainages. Je m'arrêterai d'abord sur le formalisme de ces parrainages. Il est regrettable que leur transmission électronique, prévue pourtant depuis plusieurs années, soit repoussée après la prochaine élection.

Quand on voit- et c'est à saluer ! -que le service des impôts a réussi à généraliser la numérisation des déclarations de revenus, il est regrettable qu'aucune solution n'ait été trouvée pour s'assurer de l'effectivité d'une décision vieille de cinq ans.

ma part attirer votre attention sur un sujet trop longtemps oublié, le vote des détenus. Fait rare, je citerai notre président Emmanuel Macron qui, alors candidat, avait rappelé : « On a essayé de m'expliquer pourquoi des détenus ne pouvaient pas voter. Je n'ai pas compris. Il semblerait que ce soit le seul endroit de la République où l'on ne sache pas organiser le vote par correspondance ni l'organisation d'un bureau. » Les autorisations de sortie pour aller voter sont peu nombreuses. Malgré le succès relatif de l'établissement de bureaux de vote lors des élections européennes, il a été décidé de ne pas renouveler l'expérience pour se concentrer sur le seul vote par correspondance.

Ce texte prévoit aussi que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques mette en oeuvre, à titre expérimental, un téléservice permettant l'édition et la délivrance de reçus pour chaque don versé à un candidat. Elle devra aussi, toujours à titre expérimental, mettre en place un téléservice pour recevoir de manière dématérialisée les comptes de campagne des candidats à l'élection présidentielle. J'espère que cette simplification numérique bénéficiera des mêmes critères de sécurité qui justifient le non-recours à la dématérialisation des parrainages. Toujours en termes de simplification, les électeurs dits « Français de l'étranger » pourront désormais avoir recours au vote par procuration sans avoir besoin de justifier d'un empêchement. Comment justifier que ce changement ne s'applique qu'aux Français de l'étranger ? Cette interrogation est à l'origine d'un amendement d'appel que j'ai présenté devant la commission. Si cette règle, qui revient à considérer que le vote par procuration est une modalité et non une exception, s'applique à tous, d'autres aménagements sont à prévoir. Ils devront tenir compte des enseignements tirés du dévoiement passé de ce vote peu sincère. Enfin, notre commission a choisi d'apporter davantage de lisibilité aux sondages publiés. Dans une période où chacun pense pouvoir commenter et interpréter des chiffres diffusés de manière brute au mieux, de manière orientée le plus souvent, au nom d'une transparence dévoyée,

Cerise sur le gâteau : que dire de l'amendement de dernière minute du Gouvernement ? Au-delà du processus et de son dépôt tardif, au-delà des risques et des inconvénients non évalués par le Conseil d'État, au-delà de l'absence de volonté réelle de faire évoluer nos processus électoraux, je vous incite, mes chers collègues, à vous pencher sur l'étiologie de la décision ayant conduit au dépôt de cet amendement.

en gouvernant seul, hors du cadre régulier prévu par notre démocratie, se permet en quelque sorte d'échapper aux électeurs. Notre système est à bout de souffle, notre démocratie fragilisée, pas seulement en raison des mesures restrictives prises au nom de la lutte contre la pandémie. Cette tiédeur dans l'établissement de nouveaux contours pour l'élection qui est au coeur de notre système n'est pas de bon goût, en tout cas pas de notre goût. C'est pourquoi le groupe GEST n'approuvera pas ce projet de loi.

Sous votre présidence, monsieur le sénateur Buffet, les membres de votre commission ont introduit seize amendements. D'autres seront discutés cet après-midi. Comme cela a été rappelé, contrairement aux autres scrutins électoraux, les règles applicables à l'élection présidentielle relèvent de la loi organique.

pour la première fois, de la « déterritorialisation » des procurations, prévue par la loi Engagement et proximité de 2019 à la campagne officielle, dont le calendrier serait élevé au rang de disposition organique. Sa durée resterait cependant inchangée : elle commencerait toujours le deuxième lundi précédant le scrutin pour s'achever la veille de l'élection. été ajoutées en commission : la sécurisation du vote par procuration des majeurs protégés dans les outre-mer, et l'obligation faite aux instituts de sondage de publier leurs marges d'erreur. En outre, le texte comporte un certain nombre de dispositions telles que, à l'article 1, les opérations préparatoires au scrutin. Il sécurise notamment, à titre subsidiaire, la composition des commissions de contrôle qui veillent à la régularité des listes électorales des Français de l'étranger. D'autres mesures figurant à l'article 4 intéressent spécifiquement les 3,5 millions de Françaises et de Français vivant à l'étranger. Le projet de loi organique précise aussi que la création d'une procédure dématérialisée de transmission des parrainages sera reportée à 2027 au plus tard, en raison du retard pris dans la mise en place de moyens d'identification électronique offrant un niveau de garantie élevé. La commission des lois a actualisé la liste des parrains, tirant les conséquences des récentes réformes territoriales, et en ajoutant les présidents des conseils consulaires des Français de l'étranger. Nous y sommes bien entendu favorables. L'article 2 porte sur les règles visant à encadrer le financement de la campagne. Le texte prévoit d'imposer la dématérialisation des reçus-dons délivrés aux personnes physiques ayant consenti des dons, ainsi que du dépôt des comptes de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Alors que le report des élections régionales et départementales de mars à juin 2021 a pour conséquence le chevauchement des périodes de campagne financière des élections locales et de l'élection présidentielle, vous avez reculé au 1juillet 2021 le début de cette période pour l'élection présidentielle. Le texte prévoit que le vote par correspondance papier soit ouvert aux détenus, en complément du vote par procuration et des permissions qu'ils peuvent solliciter pour se rendre jusqu'à leur bureau de vote. Sur environ 55 000 détenus ayant conservé leurs droits civiques, seuls 2 % ont participé à l'élection présidentielle de 2017. Il s'agit de réduire cette abstention massive. Par ailleurs, mes chers collègues, au-delà des suspicions, des polémiques et des avis radicaux sur la chance que pourrait représenter le vote par anticipation, qui- nous l'avons bien compris -ne sera pas adoptée, je souhaite revenir sur la proposition du sénateur Mouiller. Nous partageons largement l'objectif que celui-ci vise, puisqu'il tend à donner un accès plein et entier à l'information sur tous les candidats et leur programme à tous les Français, sans omettre les personnes en situation de handicap. Ainsi, en 2022, tous les candidats à l'élection présidentielle seront soumis à de nouvelles obligations en matière d'accessibilité de leur campagne. Ils devront tenir compte des différentes formes de handicap et de la diversité des supports de communication.

nous pouvons considérer que ce projet de loi organique inaugure le cycle cérémoniel inhérent à la VRépublique. D'abord, il procède à ce qu'il est convenu d'appeler un « toilettage » électoral, tant nécessaire qu'habituel en raison du caractère organique de la loi de 1962, et sur lequel il n'y a pas lieu de s'attarder. Il répond en effet au besoin de coordination et d'actualisation des renvois opérés par la loi du 6 novembre 1962 vers le code électoral. Le texte comporte aussi certaines dispositions techniques attendues, par exemple celle qui tend à imposer la dématérialisation des reçus-dons, que le Sénat a eu la sagesse de restreindre à un dispositif expérimental plutôt que de la pérenniser sans recul. Mais le projet de loi que nous discutons pourrait aussi comporter certaines innovations majeures au sujet desquelles il faut faire preuve de vigilance. Par exemple, nous allons devoir examiner un amendement du Gouvernement sur le vote par anticipation. Par ce mécanisme, les électeurs pourraient être amenés à voter dans une autre commune plusieurs jours avant le dimanche traditionnel du scrutin. Cette disposition appelle deux remarques. D'abord, du point de vue de la procédure parlementaire, nous nous inquiétons de cet usage toujours plus fréquent du droit d'amendement, qui conduit à introduire, souvent de manière inattendue, des éléments majeurs de réforme dans notre législation. Nous pourrions attendre qu'ils soient discutés, notamment à l'occasion de l'examen des rapports en commission, c'est-à-dire avec davantage de temps, de recul et de profondeur. Or tel n'est pas le cas : par ce biais, les échanges sont réduits et les travaux moins éclairés. Ensuite, s'agissant du fond, il s'agit d'un mécanisme étonnant qui conduit à désacraliser les dimanches de scrutin. Cela pose notamment la question de son articulation avec la campagne, habituellement suspendue la veille du scrutin. Qu'en sera-t-il avec ces votes anticipés ? Qu'adviendra-t-il également du débat organisé entre les deux tours ? Certains pourront-ils voter avant qu'il ait lieu ? Je ne doute pas que des solutions juridiques et techniques pourront être apportées, mais elles ne lèveront pas les interrogations pratiques et politiques sur le sens du résultat d'un scrutin étalé dans le temps. Enfin, comme avant chaque scrutin, la question du mode de désignation des candidats se posera. Certains voudraient se positionner en faveur d'une réforme abaissant le nombre de parrainages habituel au bénéfice d'un système hybride, sur le modèle d'une pétition nécessitant un « parrainage citoyen En plus de douter des bienfaits d'un tel système, j'aimerais dire un mot de la portée symbolique que pourrait avoir ce changement. Nos élus locaux ne sont pas des élus d'une espèce qu'il faut dévaluer. Eux aussi incarnent la démocratie J'ajoute que leur démocratie s'exerce le plus souvent loin du populisme médiatique, au contact du réel, sur le terrain. Pour ces raisons, notre République doit maintenir leur rôle historique à tous les niveaux. Et, plutôt que de vouloir les écarter progressivement des institutions étatiques, rappelons-nous le lien privilégié que ces élus ont toujours entretenu avec la Nation et ses territoires. Rappelons-nous également la confiance historique qui leur est accordée depuis des décennies, et face à laquelle ils ont rarement déçu. Souvenons-nous, par exemple,

Ce tableau laisse rêveur. Nous renonçons déjà depuis plusieurs mois à ces convivialités gustatives. Alors, s'il vous plaît, mes chers collègues, n'y ajoutons pas le renoncement aux services de ceux qui parrainent localement, depuis plus d'un demi-siècle, les candidats à la plus élevée des fonctions républicaines. Aussi, vous comprendrez que ce n'est que sous réserve du sort qui sera réservé à certains amendements déposés en séance que le groupe RDSE votera en faveur de ce texte.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, ce texte met à jour des dispositions techniques et prévoit de nouveaux dispositifs pour les prochaines élections présidentielles.

L'élection présidentielle est la clé de voûte des institutions de la V République. Vous avez rappelé, monsieur le rapporteur, que l'élection présidentielle au suffrage universel direct donne des pouvoirs très forts et très singuliers au Président de la République, chef de l'État. Vous avez également rappelé comment, depuis vingt ans, la présidentialisation- je dirai même l'hyperprésidentialisation -s'est accrue. Nous assumons la dénonciation d'une pratique monarchique du pouvoir et d'un dévoiement des institutions républicaines qui, rappelons-le, se fondent sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cette présidentialisation, comme vous l'indiquiez, monsieur le rapporteur, a été précipitée par l'instauration du quinquennat et l'inversion du calendrier électoral. La dérive que nous vivons aujourd'hui exige de rendre au Parlement son pouvoir et de le rétablir comme pivot de la démocratie. Elle exige de revenir aussi vite que possible sur l'inversion du calendrier électoral. de revenir sur la durée du mandat du Président de la République. Elle exige enfin d'ouvrir un débat sur les prérogatives de ce dernier. La crise sanitaire, nous le voyons bien avec la captation du pouvoir par l'exécutif, accélère l'exigence d'une révision en profondeur de nos institutions. Oui, nous estimons qu'il faut changer

équité aux contours incertains, reposant souvent sur des sondages qui, rappelons-le, sont produits par des instituts aux mains de grands groupes privés, peu enclins à la neutralité dans le débat politique. Les sondages doivent être encadrés, limités, voire interdits durant une certaine période. Nous le voyons bien dès à présent, plus d'un an avant l'élection, certaines forces font déjà l'impasse sur le premier tour : ce sera un duel Macron-Le Pen, point barre ! La messe serait ainsi déjà dite et le pluralisme étouffé. Le système américain lui-même montre bien que la bipolarisation de la vie politique tue la démocratie à petit feu. La question de l'argent dans les campagnes présidentielles n'est abordée dans ce texte que par un biais lointain ; elle doit pourtant être posée clairement. Pour favoriser ce pluralisme si nécessaire, pour favoriser l'égalité des candidatures, il faut limiter le niveau des dépenses électorales. Nous proposerons de les abaisser significativement. Nous proposerons également d'abaisser le seuil de remboursement des frais de campagne. Vous le constatez, ces trois thématiques, parmi d'autres, comme celle qui viendra en débat sur les parrainages, sont fondamentales. Enfin, nous proposerons qu'une réflexion soit engagée sur les conditions de déroulement d'une campagne présidentielle dans les mois qui précèdent le scrutin. Le risque existe que, au moins à l'automne, nous ne soyons malheureusement pas sortis de l'épidémie, même si nous espérons toutes et tous le contraire. Comment permettre à ceux qui n'ont pas au moins accès aux médias de mener leur campagne durant une telle période ? Il faudra par exemple réfléchir à élargir le temps d'antenne longtemps avant la campagne officielle ou à créer une plateforme numérique pour ouvrir dans l'égalité les nécessaires moyens technologiques à tous. L'abstention ne se combattra pas de surcroît durant une crise sanitaire par des évolutions, voire des manipulations, techniques, comme le propose le Gouvernement par un amendement tendant à créer un droit à voter de manière anticipée. Notre groupe, comme d'ailleurs une majorité de nos collègues, est indigné, choqué, tant sur la forme que sur le fond, par la méthode du Gouvernement, méprisante, et par cette volonté permanente de remettre en cause la démocratie citoyenne par des artifices de modernité. Je rejoins ainsi les propos de M. le rapporteur. L'abstention se réduira justement par le débat, par la démocratie, par la conviction que le vote est utile. Nous ne voterons pas contre ce texte ; nous nous abstiendrons, car il est trop limité pour répondre à l'urgence d'un sursaut démocratique. La parole

et le sujet qui vous est en réalité soumis n'était pas un objet du texte initial. Je ne reviendrai pas sur les amendements ni sur la présentation technique

etc. Cela nous est présenté comme une tradition républicaine. Or j'aurais plutôt tendance à considérer qu'une vraie tradition républicaine consisterait à stabiliser les conditions de l'élection présidentielle et à ne plus toucher, sauf absolue nécessité, à la loi de 1962.

cette disposition n'avait jamais été envisagée dans le texte initial. Un point de procédure préalable : si vous rejetez tout à l'heure cet amendement n° 32, ce rejet sera définitif,

les seuls amendements susceptibles d'être adoptés après la réunion de la commission mixte paritaire doivent être soit en relation directe avec une disposition restant en discussion, soit dictés par la nécessité de respecter la Constitution,

Pour les sénateurs centristes, cet amendement est « abracadabrantesque » et source de désordre. Nous voterons donc très clairement pour son rejet. Si l'objectif est un effet de faire évoluer notre mode de votation et d'expérimenter un vote par anticipation, la raison voudrait qu'on le fasse à l'occasion d'une élection locale.

Si l'objectif était de favoriser la participation, chacun le ferait sien. Nombreux ont été les sénateurs

était d'intégrer l'hypothèse d'un maintien de la pandémie en mai 2022, l'idée de concentrer le vote par anticipation sur une centaine de bureaux semblerait plutôt aboutir à un résultat défavorable sur le plan sanitaire. peu dire que je ne vois pas de fondement sérieux à cet amendement n° 32. Au-delà de la forme très inélégante- son apparition subite, sans aucun aucun préalable, sans aucune concertation, sans aucun travail, sans aucune évaluation, sans aucune réflexion commune et, finalement, alors que c'est toujours nécessaire dans un exercice démocratique, sans aucune forme de maturation -, les motifs de son rejet sont multiples. Je retiendrai essentiellement deux motifs de rejet de cet amendement. Le premier, c'est la rupture du lien entre le vote et un territoire, cette alchimie qui a habitué nos concitoyens à se retrouver au même endroit

la défiance de notre société en général, la société française de 2021 étant un concentré de défiance. Au risque d'une formule un peu excessive, je crois même qu'on pourrait dire que notre pays est malade de cette défiance. L'amendement n° 32 ajoute encore de la défiance, tant les machines à voter ne sont pas intégrées à notre culture démocratique. Le vote relève de différentes composantes : il y a une dimension culturelle ; il y a une forme de rituel républicain, de rituel individuel, de rituel dans sa dimension collective. Je ne crois pas que, à l'occasion de l'élection présidentielle, il soit sage d'y porter atteinte. Finalement, l'amendement n° 32 a un mérite : en lien avec les propositions de loi sur l'introduction de la proportionnelle ou d'une part de proportionnelle, il souligne le malaise institutionnel résultant de la concentration des pouvoirs entre les mains de l'exécutif.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, en 1959, le juriste Georges Burdeau se demandait où était incarné le pouvoir dans la Constitution de la V République. Il concluait tout simplement que ce pouvoir,

Cela veut dire tout simplement que la révision de 1962 n'a pas été un changement de nature, mais un changement de degré par rapport au pouvoir donné au Président de la République, un virage institutionnel. C'est ce qui fait que nous nous retrouvons là aujourd'hui, tout simplement parce que l'élection du Président de la République ne figure pas dans le code électoral. D'où cet exercice ritualisé que nous exécutons tous les cinq ans. La vraie question est : « Faut-il continuer à procéder à ce rituel à un moment où nous faisons face à des circonstances exceptionnelles ? C'est ce que propose la majorité sénatoriale, c'est ce que proposait l'exécutif avant son de mardi dernier. En réalité, même un texte technique reste un texte politique,

Cela voudrait dire aussi que la sacralisation de l'élection présidentielle ne nous permet pas de procéder à sa modernisation. Or, me semble-t-il, il faut se garder des idoles, parce que, justement, en adoptant cette attitude, on en vient à intérioriser l'importance définitive de cette élection. Le texte qui nous avait été proposé initialement était un texte de réglages, sans ambition majeure : une actualisation nécessaire avant chaque scrutin,

de la commission des lois : la convocation des électeurs par décret simple, l'actualisation de la liste des parrains, le caractère expérimental de la dématérialisation des comptes de campagne et des « reçus-dons », l'obligation de publication des marges d'erreur par les instituts de sondage- après l'adoption d'un amendement de Jean-Pierre Sueur -,

pour le dire simplement, nous avons tout essayé : le vote par correspondance en 2022, le vote par correspondance par expérimentation, le vote par correspondance en 2027 Nous avons aussi tenté de mettre en place un vote par anticipation, non pas au sens où l'entend le Gouvernement, mais étendant la période de vote au vendredi, au samedi et au dimanche.

Arrive l'amendement du Gouvernement, qui a un avantage : faire l'unanimité contre lui. Comment tuer une bonne idée potentielle ? Eh bien ! je vais vous donner la réponse : comme ça Sur la méthode, cet amendement est tellement bon qu'il n'a besoin ni d'étude d'impact, ni d'un avis du Conseil d'État, ni de concertation. Pour le coup, le Gouvernement a été vraiment « en marche » contre sa majorité à l'Assemblée nationale. Les délais ne laissent aucune place à la réflexion. Pas d'analyse, pas d'expertise. Il est vrai que la force immanente de ce gouvernement est telle qu'il n'en a pas besoin ... Cet amendement tombe du ciel, dans toute sa verticalité jupitérienne, en catimini, à l'issue de la navette parlementaire. Bref, c'est parfait ! Sur le fond, nous avons le sentiment d'une improvisation, d'un grand flou, et quand c'est flou, vous connaissez la suite amendement est structurellement défectueux : il modifie la question de l'anticipation, la question de la déterritorialisation et l'extension du recours aux machines à voter. Sur l'anticipation du vote, la date est arrêtée par décret. On est tranquilles ... De nouveau, les parlementaires Sur la déterritorialisation, cela a déjà été dit, quelles sont les modalités de mise à jour des listes d'émargement en ce qui concerne le double vote ? Faudrait-il en fait aider un électorat mobile, bien intégré socialement ? Suivez mon regard ! ... Sur l'extension du recours aux machines à voter, le moratoire

Sur la technique des machines à voter en tant que telle, il y a eu de multiples travaux en la matière. Il existe une certitude : un rapport du HackingVillage de 2019 souligne qu'aucune machine à voter

C'est en tout cas la traduction que Gérald Darmanin en a faite devant le rapporteur, le même Gérald Darmanin qui nous jurait la main sur le coeur que, en dehors du vote à l'urne, il n'y avait pas de salut ! Si cet engagement était aussi important, alors pourquoi avoir balayé l'ensemble des propositions du revers de la main ? serait là la manifestation d'une volonté de moderniser le droit électoral et d'anticiper. Stéphane Séjourné, qui a la particularité d'être conseiller spécial du Président et eurodéputé LREM, nous explique doctement que le sujet, c'est la modernisation de notre démocratie. Christophe Castaner, le responsable de la majorité écrasée dont je parlais tout à l'heure, nous explique que la proposition, au sens où on l'entend, serait effectivement une réponse au contexte sanitaire.

En définitive, et on le sait bien, cet amendement n'a pas vocation à aboutir. La vraie difficulté, c'est que les Français retiendront de cette séquence inopportune le sentiment d'un tripatouillage politique, même si ce n'était pas vraiment l'intention.

nous entamons donc l'examen de ce projet de loi organique relatif à l'élection du Président de la République, texte indéniablement important pour le bon déroulement de l'élection la plus centrale des institutions de la V République,

nécessaire au regard des évolutions du code électoral depuis le dernier scrutin. C'est ainsi que ce texte organique détermine un certain nombre des paramètres nécessaires au déroulement de l'élection modalités de convocation des électeurs, règles applicables aux parrainages, au vote des détenus, aux comptes de campagne, aux procurations ou encore aux Français de l'étranger. Je ne reviendrai pas en détail sur ces points, qui n'ont, pour la plupart, pas fait l'objet de difficultés insurmontables. Les travaux de notre commission des lois ont volontiers suivi cette logique de toilettage. Pour cela, elle a procédé à un certain nombre d'améliorations de nature à faciliter et à moderniser le déroulement de la campagne et du scrutin. Il en est ainsi de la publication en des comptes de campagne, utile gage de transparence du processus électoral, ou encore de l'ouverture des parrainages aux vice-présidents des conseils consulaires. Cette dernière mesure, à laquelle, vous l'imaginez, je suis assez sensible, est réclamée depuis 2015 par le Sénat. Bien qu'elle ne concerne que 152 vice-présidents et- bientôt -présidents de conseil consulaire, elle constitue la reconnaissance de leur engagement au service de la démocratie, y compris hors de nos frontières. suite du report des élections départementales et régionales, que nous avons voté en début de semaine, il a paru judicieux à la commission de prendre les mesures s'imposant afin d'éviter que ne se chevauchent les périodes des comptes de campagne de ces scrutins et de l'élection présidentielle. Si mon intervention se limitait à ces considérations « techniques », elle passerait à côté de ce qui est devenu, par la force des choses et, surtout, des choix de l'exécutif, le point le plus saillant de l'examen du projet de loi organique je parle bien évidemment, mes chers collègues, de la question du vote par anticipation au moyen de machines à voter. Par un amendement présenté ce mardi, à la veille de la réunion de la commission des lois sur les amendements extérieurs, le Gouvernement a proposé d'intégrer dans la loi organique un dispositif complexe et inédit instaurant le vote par anticipation à la présidentielle de 2022. Ce dispositif, qui, forcément, ne figure ni dans l'étude d'impact ni dans l'avis du Conseil d'État, nous arrive en queue de processus législatif, pratiquement au stade de la commission mixte paritaire. Même si nous sommes malheureusement accoutumés à ces coups de théâtre du troisième acte, cela interroge tout de même sur l'approche du débat parlementaire qu'a le Gouvernement. Le fond de l'amendement n'en soulève pas moins des interrogations il s'agirait de permettre aux électeurs de voter le mercredi précédant la date normale du scrutin dans une liste de communes- probablement les chefs-lieux de département -au moyen de machines à voter électroniques. D'une part, avons-nous les moyens de déployer, sous un an, sans expérimentation préalable ni travaux en profondeur, des machines à voter qui garantissent toutes les conditions de sécurité technique et procédurale ? Peut-être au prix d'un effort logistique considérable avec un énorme risque potentiel D'autre part, et de manière plus grave encore, cet amendement pose des questions d'ordre démocratique. Privilégier certaines grandes communes découle peut-être de considérations logistiques, mais revient à engendrer une rupture d'égalité devant le vote, certaines personnes vivant loin de ces villes.

Le même problème, à une échelle moindre, se retrouvera dans de nombreux territoires ruraux de l'Hexagone. Dans le contexte politique actuel, cela relèverait d'un bricolage susceptible d'engendrer des suspicions sur les objectifs du Gouvernement et d'endommager, ce faisant, la sincérité du scrutin. En outre, le vote anticipé pose la question du changement de vote. Que se passerait-il si les événements faisaient que l'électeur décide de modifier son choix entre le mercredi et la fin de la semaine ? Pourrait-il voter de nouveau et remplacer son ancien vote ? Ou serait-il contraint de s'en tenir à un choix qui n'est déjà plus le sien ? Je n'entrerai même pas dans le détail de la critique qui peut être faite du principe du recours aux machines. Cette pratique existe effectivement dans certaines communes, mais n'oublions pas que ce principe fait l'objet, depuis la présidentielle de 2007, d'un moratoire en raison des risques de fraude identifiés par le Conseil constitutionnel lui-même. Comme ont pu le relever les membres de la mission d'information sur le vote à distance mise en place par la commission des lois à la fin de l'année dernière, l'éventuel intérêt théorique et à moyen terme d'une évolution du droit électoral ne signifie pas qu'elle doive s'appliquer immédiatement et sans préparation, quand l'enjeu est l'élection du Président de la République. J'espère donc que le Gouvernement aura la sagesse de reconnaître l'inopportunité de cet amendement et le retirera. le groupe Les Républicains votera donc le texte du projet de loi organique dans sa rédaction issue des travaux de la commission des lois. La discussion

Mme Éliane Assassi. L'état d'urgence sanitaire, nous l'avons dit et répété, porte une atteinte considérable aux libertés publiques et aux libertés démocratiques. Logiquement, le calendrier électoral et le processus électoral sont bousculés, comme on l'a vu avec les élections municipales, les élections régionales et départementales. Cela dit, reporter l'élection présidentielle nécessiterait une révision de la Constitution qui n'apparaît ni réaliste ni souhaitable. L'élection présidentielle aura donc bien lieu à la date prévue.

D'ici à ce que l'élection présidentielle batte son plein, nous pouvons raisonnablement espérer que les conditions sanitaires permettent aux candidats de faire campagne. Par ailleurs- M. le rapporteur l'a indiqué -, l'article 58 de la Constitution confère au Conseil constitutionnel une compétence générale qui concerne l'élection présidentielle. Le Conseil constitutionnel intervient de manière déterminante tout au long du processus électoral et tout particulièrement pour l'élection présidentielle. Il est notamment consulté par le Gouvernement sur l'organisation des élections et avisé sans délai de toutes les mesures

Certes, des garanties existent depuis la loi du 11 février 2005 pour l'accès des personnes handicapées aux bureaux de vote et aux opérations de vote. En revanche, comme le relevait dès 2014 le rapport Orliac-Gourault, les règles d'accessibilité ne s'appliquent pas aux « phases préalables au scrutin lui-même, qu'il s'agisse de la campagne officielle ou de la campagne " officieuse ", la plus longue dans les faits et au cours de laquelle interviennent les principales actions d'information ». Or l'exercice effectif du droit de vote suppose un accès plein et entier à l'information sur tous les candidats et leur programme. Le Défenseur des droits avait interpellé à ce sujet les candidats à l'élection présidentielle de 2017, constatant une grande hétérogénéité de pratiques. Il n'est pas acceptable que les campagnes électorales, largement financées par l'impôt, ne soient pas accessibles à l'ensemble de nos concitoyens en dépit des moyens techniques qui existent aujourd'hui. Cet amendement vise donc à inscrire dans la loi du 6 novembre 1962 une obligation pour les candidats à l'élection présidentielle de veiller à l'accessibilité de leurs moyens de propagande électorale aux personnes handicapées.

un vide juridique persiste : aucun cadre n'assure l'accessibilité de la campagne elle-même. Vous proposez d'aller beaucoup plus loin en inscrivant dans la loi l'obligation pour les candidats de veiller à l'accessibilité de leur propagande électorale. C'est un sujet difficile à appréhender, notamment en raison de la pluralité des formes de handicap et de la diversité des supports. Mais il paraît pleinement légitime

de déposer une seconde profession de foi en langage dit « facile à lire et à comprendre » lors des élections européennes de 2019. La même mesure sera prise pour la prochaine élection présidentielle

ainsi intelligibles pour l'ensemble des citoyens. En outre, une mission interministérielle va permettre de dresser le bilan du recouvrement du droit de vote pour l'ensemble des majeurs sous tutelle et d'évaluer

le scrutin présidentiel a toujours lieu pendant les vacances de Pâques, au moins pour une partie du territoire, pour une raison très simple : c'est que le président Pompidou est décédé le 2 avril 1974. Depuis lors, le premier tour de l'élection présidentielle a lieu au mois d'avril

Éric Kerrouche. Cet amendement vise à dissocier plus nettement la date de la publication de la liste des candidats et le début de la campagne officielle. Cette distinction nous paraît utile et importante.

modification apportée à la loi organique de 2016 permettant une publication au fil de l'eau de la liste des parrains. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel a dressé un bilan satisfaisant de cette procédure pour l'élection de 2017.

de l'ouverture de la campagne. La différence entre ces deux périodes d'équité est ténue : la seconde est dite « renforcée », dans la mesure où l'accès équitable au temps d'antenne doit se faire « dans des conditions de programmation comparables », c'est-à-dire suivant une répartition équitable, tenant compte des tranches horaires et de l'exposition des émissions de télévision. La période d'équité au sens large est donc longue : ainsi, lors de la dernière élection présidentielle, elle avait commencé le 1 février 2017. D'ailleurs, personne à l'époque n'avait appelé de ses voeux un allongement supplémentaire. Les dispositions actuelles ne présentent, à notre sens, pas de difficulté d'application. le Gouvernement est défavorable à ces amendements. Au reste, s'il fallait faire évoluer les règles en la matière, le travail à mener serait plutôt de nature réglementaire : c'est en effet l'article 7 du décret de 2001 qui encadre à l'heure actuelle les modalités de publication de la liste des candidats.

d'inaugurer les chrysanthèmes, comme on le disait sous les IIIet IV Républiques, de façon peut-être un peu caricaturale d'ailleurs. Le mode de décision a lui aussi évolué : ce ne sont plus les parlementaires, mais les Français, qui désignent le Président de la République depuis 1962. Les conditions d'éligibilité ont également évolué

Rappelons tout de même que le Président de la République française est le chef de l'État ; il est maître de la diplomatie et des armées ; il dispose du feu nucléaire ; il peut dissoudre l'Assemblée nationale ; il nomme le Premier ministre ; il a le droit de grâce- j'en passe et des meilleures.

du mode de parrainage pour l'élection du Président de la République. Le système actuel apparaît de moins en moins légitime aux yeux des citoyens, qui sont écartés de cette phase de préqualification au profit d'élus, qui eux-mêmes subissent un peu trop la pression de cette compétition.

Ce second seuil est celui qui était recommandé par la commission de rénovation et de déontologie de la vie publique. Elle le jugeait à la fois suffisamment élevé, pour limiter le risque d'émiettement des sans l'être trop, pour ne pas exclure des candidats se réclamant d'un courant politique représentatif. L'introduction des parrainages citoyens autoriserait, en contrepartie, une diminution du nombre de parrainages d'élus : ainsi, elle limiterait la pression s'exerçant

Il considère que le législateur ne saurait prévoir d'inéligibilités que dans la mesure nécessaire au respect du principe d'égalité devant le suffrage et à la préservation de

Au-delà des fraudes et des risques d'erreur, les temps d'acheminement et de contrôle sont incompatibles avec les délais prévus par la Constitution, notamment en cas de vacance ou d'empêchement définitif.

ne disqualifie pas un candidat à l'élection présidentielle, bien au contraire. Par ailleurs, subordonner l'éligibilité au scrutin présidentiel à la détention d'un mandat électif,

que la solution actuelle est la bonne, et donc écarter de fait les citoyens de cette première phase, ne nous semble pas

de publication de la liste des candidats. Ce principe d'égalité s'imposerait ainsi près d'un mois avant le premier tour, tour, introduisant une certaine rigidité qui conduirait inévitablement les médias à réduire leur couverture de la campagne présidentielle. C'est un phénomène que nous avons déjà pu observer avant 2016 avec cette double règle

le CSA doit veiller à tout moment au pluralisme de l'information, ce qui implique une forme d'équité dans la présentation et dans l'accès à l'antenne des formations politiques

Il n'en demeure pas moins que ce système fonctionne de manière assez convenable à l'étranger

Les élections se sont toujours tenues le dimanche pendant une journée, c'est le principe. Par ailleurs, si les services de l'État et des communes sont toujours au rendez-vous pour que les élections se déroulent au mieux, l'organisation d'une élection présidentielle n'en demeure pas moins exigeante et fait intervenir un nombre important de participants. Or les acteurs locaux et les élus avec lesquels nous avons échangé nous disent qu'il leur serait très probablement impossible de trouver suffisamment de personnes pendant trois jours successifs pour assurer les missions

pour les candidats du premier tour et de 33 % pour les candidats présents au second tour. S'agissant de votre second objectif, qui est d'ouvrir plus largement le droit au remboursement maximal, à savoir 47,5

des donateurs aux candidats à l'élection présidentielle n'est pas publiée ; toutefois, elle est communicable à la demande, comme l'a rappelé le Conseil d'État dans sa décision du 27 mars 2015, sous réserve de l'occultation des mentions nominatives pour éviter les atteintes à la vie privée. Les impératifs de transparence sont donc bien respectés et il n'est pas dans l'intention du Gouvernement de faire évoluer la loi de 1962 sur ce point. La transparence sur l'origine des dons

présidée par Lionel Jospin : en cas de rejet du compte de campagne du candidat proclamé élu en raison d'un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement, sans préjudice, bien sûr, des poursuites pénales, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques notifie cette décision au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat, en vue d'éclairer le Parlement, afin de lui permettre d'engager, le cas échéant, en toute connaissance de cause, une procédure de destitution. Tel est l'objet du présent amendement.

que j'ai l'honneur de représenter pour vous présenter cet amendement, je voudrais rappeler le contexte, parce que je sais à quel point le dépôt de cet amendement par le Gouvernement a pu étonner, voire susciter de la colère. Plusieurs d'entre vous l'ont dit hier à l'occasion de débats, dans les médias et, aujourd'hui, lors de leurs propos liminaires.

à la fois à l'engagement du programme du Président de la République sur la numérisation et la modernisation de la démocratie et à la volonté d'un certain nombre de parlementaires de moderniser, de numériser le vote et de faire en sorte que, en 2022, on puisse élargir les conditions d'accès à la démocratie

C'est la démocratie ! Absolument, monsieur le sénateur, et il est heureux qu'il en soit ainsi. J'en viens à la présentation de l'amendement. Les élections sont organisées avec une grande rigueur grâce à la participation active des maires, des équipes communales, de l'administration de l'État et cette rigueur se traduit par des modalités de vote simples et efficaces à l'aide d'un bulletin placé dans une enveloppe, puis dans une urne, le dimanche du scrutin ou une machine. Cette simplicité permet de réduire de manière draconienne les malfaçons, les fraudes, les polémiques, les contentieux, évite de faire peser une incertitude sur les opérations électorales et sur les résultats et permet de maintenir la confiance des citoyens dans les opérations électorales.

Bien évidemment, la méfiance de l'ensemble des citoyens français a des ressorts divers et variés, mais je voudrais poser la question du nombre d'électeurs qui auraient besoin de voter à un autre endroit que celui où ils se trouvent, qui ne se trouvent pas dans leur commune quelques jours avant le scrutin, voire le jour même du scrutin. Des

amendement ouvre la voie à une nouvelle modalité de vote, doublement originale et facilitatrice : l'électeur pourra voter dans la commune de son choix dans un délai n'excédant pas une semaine avant le scrutin. Évidemment, pour des raisons techniques et afin de sécuriser les procédures, il ne sera pas possible de voter en tout lieu

grands auteurs ont été cités : Stéphane Séjourné, Christophe Castaner, Gérald Darmanin ... En ce qui concerne le ministre de l'intérieur, je dois rappeler que, s'il s'est prononcé contre le vote

comme le scrutin électronique, soit entièrement incontestable. Des cas de fraude peuvent être relevés. » Le même a également écrit : « Nous n'avons pas besoin de cela, au moment où la légitimité des élus est attaquée. a renchéri en ces termes : « Contrairement aux Américains, les Français ont l'habitude que l'élection se tienne en une journée. Par ailleurs, il ne m'a pas semblé que le système électoral américain soit des plus incontestables, ou plus lisible que le nôtre. Je m'interroge d'ailleurs sur les volontés d'américaniser notre système institutionnel. » Je tiens l'ensemble de ces déclarations à votre disposition,

ces difficultés, notamment l'interrogation sur la fiabilité de ces machines. Or c'est le Conseil constitutionnel qui, dans sa décision de 2008, a relevé un problème de fiabilité, notamment lors des élections législatives de 2007.

vote. Certes, il faut moderniser notre vie démocratique, mais avec une certaine prudence et en concertation avec les forces politiques du pays et les élus locaux, à l'instar de ce que nous avons fait pour le report des élections régionales et départementales.

en période de crise sanitaire. Oui, nous sommes en France, mais sachons regarder un peu plus loin : nous aurions pu améliorer la proposition faite, s'agissant de l'usage des machines à voter comme du renforcement de la sécurité du scrutin, afin de garantir des résultats légitimes et incontestables. Le groupe RDPI votera tout de même cet amendement.

l'on répondra à l'envie des gens. Oui, les gens ont envie de participer au débat politique ; ils ont envie d'échanges. La vie est tellement compliquée : ils ont envie

Madame la ministre, vous avez revendiqué la « modernisation » comme étant la motivation du Gouvernement.

de modifier le texte du Gouvernement ? Belle modernisation ! Est-il moderne de modifier substantiellement le code électoral sans prendre l'avis du Conseil d'État ? Est-il moderne de présenter de présenter un tel amendement, qui concerne l'organisation de notre vie politique, sans avoir pris la précaution d'une concertation avec l'ensemble des forces politiques de ce pays

aujourd'hui au Sénat, un amendement qui ne règle pas toutes les questions fondamentales soulevées par la réforme que vous mettez en oeuvre, au point que l'on peut se demander s'il ne serait pas frappé, comme les juristes le disent, d'incompétence négative ? Vous voulez avoir les mains libres, comme d'habitude. Vous voulez tout régler par décret, comme d'habitude. Vous arrivez avec un texte qui est plein de lacunes, de failles et qui n'a pas été étudié sérieusement.

sur la sincérité du vote. Vous allez faire voter des Français alors que la campagne présidentielle est en passe d'atteindre son pic, dans les deux ou trois derniers jours de la campagne. Il y aura des électeurs qui n'auront pas tout vu et qui se seront quand même prononcés.

rapidement la situation pour avoir une démocratie stabilisée. C'est le moins que l'on puisse faire vis-à-vis des électeurs si l'on veut qu'ils aillent voter.

Le scrutin est ouvert.

La prison, comme lieu d'exécution de la peine, a pour objet la protection de la société, mais également la réinsertion du délinquant. Comment envisager une réinsertion des personnes exclues de fait, et non de droit, de la participation à la vie citoyenne que constitue le moment fort des élections ? Ce projet organique, dans la droite ligne de la loi Engagement et proximité, prévoit la possibilité pour les prisonniers, en plus des mesures déjà prises pour leur inscription sur les listes électorales, les votes par procuration et les permissions de sortie, de participer à la prochaine élection présidentielle le vote par correspondance. À défaut pour cette élection de l'établissement de bureaux de vote au sein des prisons, comme cela sera suggéré dans un amendement dont nous allons discuter ultérieurement, la possibilité de voter par correspondance est déjà une avancée qui ne saurait être freinée.

Les démarches peuvent se révéler longues et parfois compliquées pour ces publics fragilisés. Il est important d'assurer au mieux les conditions de leur inscription sur les listes électorales et les modalités de vote par correspondance. L'amendement n° 19

à l'expérimentation d'un dispositif de vote par correspondance. Alors que, d'habitude, leur participation aux échéances électorales est basse- 2 % à l'élection présidentielle de 2017 et 1 % aux élections législatives de la même année -, elle a été de 8 %. a été de 8 %. Ce chiffre montre qu'il y a une volonté démocratique au sein des établissements pénitentiaires et que, lorsque l'on met en place des dispositifs allant vers une amélioration de l'accès au droit de vote, les détenus s'en saisissent. Les seules possibilités actuelles de solliciter une sortie pour aller voter ou de voter par procuration sont très complexes à mettre en oeuvre. Le présent texte prévoit le vote par correspondance des détenus pour la prochaine élection présidentielle.

préconisons existent déjà dans des pays comme le Danemark ou la Pologne, qui installent des bureaux de vote dans les prisons. Nous pouvons en faire autant. Notre amendement s'inscrit dans cette logique de permettre à chacun d'exercer ce droit, mais également de lutter contre l'abstention de personnes en situation précaire.

Comment faire, par exemple, lorsqu'un détenu sort de prison très peu de temps avant le scrutin et qu'il n'a pas le temps de changer de liste électorale ?

dans la sécurité du scrutin. Comment organiser un scrutin le dimanche à l'intérieur de ces établissements, alors que normalement le nombre de surveillants y est inférieur le week-end ?

Le Gouvernement comprend les raisons pour lesquelles cet amendement a été déposé et adopté. Le report des élections régionales et départementales de mars à juin 2021 a pour conséquence de faire se chevaucher les périodes de campagne financière des dépenses, d'une part, des élections départementales et régionales et, d'une part, de l'élection présidentielle. Conscient des difficultés que cette superposition pourrait faire naître, le Gouvernement a interrogé le Conseil d'État sur l'opportunité d'un tel raccourcissement. Éclairé par son avis, le Gouvernement propose de s'en tenir au droit commun. Tout d'abord, la superposition des périodes de contrôle afférentes à des campagnes électorales est habituelle. Elle est même systématique en ce qui concerne le scrutin présidentiel et les élections législatives. Il est fréquent qu'une même personne soit candidate à ces deux élections. Par ailleurs, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a assuré pouvoir clairement distinguer les dépenses qu'un candidat aux deux élections différentes pourrait engager. Ensuite, le raccourcissement de la période applicable à l'élection présidentielle retarderait de trois mois la mise en oeuvre du contrôle du recueil des fonds, ce qui conduirait à minorer l'encadrement des dépenses et des recettes, et donc le contrôle réalisé par la Commission. Enfin, une réduction de trois mois de la période de computation des dépenses devrait en toute logique s'accompagner d'une diminution du plafond des dépenses qu'un candidat peut engager, ce que ne prévoit pas la disposition adoptée

Nous avons auditionné le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques : les critères ne sont pas clairs

pour le début de la campagne officielle, précisant que la plateforme ne serait ouverte qu'après publication de la liste des candidats officiels à la présidence de la République. Je retirerai donc cet amendement si le Gouvernement confirme bel et bien ses propos.

avec les référés d'heure à heure que connaît bien le président de la commission des lois n'est même pas assurée. Notre collègue a donc rédigé un amendement visant à prévoir une voie de recours spécifique inscrite dans nos dispositions électorales au cas où un retrait de compte par une plateforme numérique serait susceptible d'impacter le déroulement de l'élection présidentielle ou d'une autre élection dans notre pays.

le contenu du droit d'accès à ces plateformes, les titulaires de ce droit et ses limites. Il faudrait enfin déterminer la compensation offerte aux opérateurs privés qui seraient soumis à cette nouvelle charge de service public, faute de quoi le dispositif serait contraire au principe d'égalité devant les charges publiques. C'est seulement que

l'adoption de la loi organique du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information. Ce texte vise, dans le cadre de l'élection présidentielle, à contrer la diffusion massive et rapide de fausses nouvelles les outils numériques, notamment les opérateurs de plateforme. Il prévoit, pour la période de campagne électorale, une obligation de transparence des plateformes, une obligation de signalement une action judiciaire en référé pour faire cesser rapidement la circulation de fausses nouvelles. C'est le juge des référés qui qualifiera la fausse nouvelle, selon la définition de la loi de 1881. Ces dispositions sont encore récentes. Elles visent à doter la lutte contre les fausses nouvelles d'un cadre juridique adapté en donnant tout son rôle au juge dans le cadre de la liberté d'expression. C'est principalement le souci de préserver la campagne électorale présidentielle de potentielles tentatives d'influence qui a motivé

L'ouverture des enveloppes avant le scrutin pourrait faire l'objet de certaines critiques, même en présence de magistrats indépendants. La mission d'information proposait effectivement

volontaires de voter par correspondance, ce qui constituerait une forme de rupture d'égalité devant le suffrage entre les électeurs de ces communes volontaires et les autres. Pour toutes ces raisons, j'émets un avis défavorable sur ces trois amendements.

travers cet amendement, nous proposons d'interdire les sondages portant sur le second tour de l'élection présidentielle avant même que le premier tour ne se soit déroulé. C'est lors de ce premier tour que s'organise réellement la démocratie électorale du pays. C'est le moment de l'expression pluraliste et du débat d'idées. Brûler l'étape du premier tour, ce que font allègrement les instituts de sondage qui oeuvrent de fait pour la bipolarisation de la vie politique, c'est mettre en péril l'exercice plein et entier du suffrage universel.

le fameux scrutin majoritaire à deux tours, qui jalonne cette élection, qui engendre une certaine forme de bipolarisation de l'élection. Pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, j'émettrai un avis défavorable

me paraît un enjeu crucial pour une démocratie équilibrée. L'inertie ou la dynamique des intentions de vote dont ils sont la cause ou l'objet, le des publications à un moment qui peut être téléguidé selon divers intérêts : tous ces éléments doivent nous amener à être très prudents

En ne permettant qu'à ces derniers de se soustraire à une attestation sur l'honneur justifiant « l'impossibilité de se rendre au bureau le jour du vote », le déséquilibre avec les électeurs résidant en France me paraît important. Aussi, il semble nécessaire d'établir une règle claire dans le vote par procuration : soit c'est un droit pour le citoyen, auquel cas aucune justification pour y avoir recours ne devrait être requise quel que soit l'endroit du vote, soit c'est une exception dans l'exercice du droit de vote, auquel cas une justification de l'impossibilité de se rendre au bureau de vote est nécessaire pour l'ensemble des électeurs.

à la réglementation. Nous proposons de nous saisir de ces nouvelles opportunités de communication en créant une plateforme numérique publique commune à l'ensemble des candidats. Cet outil numérique servirait l'intérêt général en donnant un accès égal aux candidats, avec par exemple un site internet et une application mobile pour y faire campagne. Parce que les candidats n'ont pas les mêmes moyens, une telle plateforme permettrait de résorber ces inégalités et de favoriser le pluralisme. La mobilisation de ces outils s'inscrit aussi dans la lutte contre l'abstention électorale en touchant un public plus large comme les jeunes, qui sont particulièrement connectés, mais aussi particulièrement en recul dans la participation électorale. Quel est l'avis de la commission ? Cet

modifié, l'ensemble du projet de loi organique, dont la commission a rédigé ainsi l'intitulé : « projet de loi organique portant diverses mesures relatives à l'élection du Président de la République ». En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public

Le scrutin est ouvert.

Le Sénat a adopté. Par courrier en date de ce jour, M. François-Noël Buffet, président de la commission des lois, demande l'inscription à l'ordre du jour de la proposition de loi tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention, sur laquelle le Gouvernement a engagé la procédure accélérée ce jour. Nous pourrions inscrire l'examen de ce texte le lundi 8 mars, à seize heures et le soir. La commission des lois se réunira pour établir son rapport et le texte le mercredi 3 mars, matin, et le délai limite pour le dépôt des amendements de séance serait fixé au lundi 8 mars à douze heures. Y a-t-il des observations ?